Merci madame la présidente, il s'agit effectivement d'une correction sur le scrutin numéro 78 du 15 janvier renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, madame Ellen qu'on nous et Mourey, qui a été compté parmi celles et ceux qui se sont abstenus lors de ce scrutin public souhaite voter contre, je vous remercie donc de bien vouloir enregistrer cette correction. Acte est donné de votre mise au point, elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l'analyse politique du scrutin concernés. alors. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales et je vais donner la parole à Monsieur Jérôme Bascher. Oui Oui bonjour madame le président, monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais appeler l'attention du ministre et il y a, a de l'ensemble du gouvernement sur la situation du Groupement hospitalier du sud de l'Oise, voilà 10 ans, ce groupement a été créé par la fusion des 2 hôpitaux de Creil et de Senlis et je m'étais exprimé à l'époque pour afin de mutualiser à 10 kilomètres d'écart, des services et d'avoir partout des choses performante plutôt d'avoir des choses moyenne à 10 kilomètres d'écart. Hélas, 1000 fois hélas tout ceci ne fonctionne pas dysfonctionne pire encore. aujourd'hui même, les urgences de Senlis, la ligne de ce mur de Senlis sont fermés. Jusque. Jusque, on ne sait pas et voilà le problème : cet été, ça avait déjà fermé en août et j'ai jusque septembre, il a fait, il fallut une grande mobilisation de l'ensemble des élus, dont moi-même, pour que celle-ci rouvre et là nous sommes dans l'expectative, alors Monsieur le ministre, que pouvez-vous nous annoncer de positif de ligne claire pour ce service d'urgence. Merci, la parole est à monsieur Adrien taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Merci beaucoup madame la la présidente, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, le Groupement hospitalier public du Sud-Ouest qui est déployée sur 2 sites distants de 15 kilomètres entre Creil et Senlis, vous l'avez rappelé fait l'objet, pour la raison que vous avez exposé une attention toute particulière de de l'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France je me permets les connaissons bien de dents salué la disponibilité à l'écart des des équipes médicales mais aussi je crois des élus de terrain qui ont été associés tous ces derniers temps, je crois au discussions réflexions qu'il y a sur la question que vous soulevez, notamment le de décembre dernier encore, je crois à l'occasion d'une visioconférence à laquelle vous avez participé alors vous le savez, en raison d'un manque de ressources médicales et en vue d'assurer les conditions optimales de prise en charge des patients et de travail des professionnels effectivement les urgences adultes du groupement ont dû être temporairement regroupées sur le site de Creil. Qui connaît le plus grand nombre de passages et qui disposent aussi du tableau du pardon du plateau technique le plus le plus important auparavant bien sûr 2 options avaient été étudiés, mais celle-ci est apparue comme la seule à même d'apporter le plus grand nombre de sécurité à à l'activité, ce regroupement a permis d'assurer la qualité et la sécurité des prises en charge, je salue les équipes qui se sont mobilisés à cette attention et je souligne la coopération avec le centres hospitalier du territoire, en particulier celui de Beauvais, ainsi que la recherche de partenariats qui a été engagée avec les professionnels de ville pour faciliter, développer l'accès aux soins non programmés, qui ne nécessitait pas recours aux urgences hospitalières problématique dont nous avons débattu à de nombreuses reprises dans cet hémicycle, dans la perspective désormais c'est votre question, et de renforcer l'effectif médical autour d'un projet médico- soignant qui soit rénové et qui soient attractifs puisque je l'évoquais, c'est un problème de ressources médicales qui expliquent la la situation actuelle, une réouverture du service d'urgences de Senlis pourrait ainsi intervenir après le recrutement de 3 à 4 médecins urgentistes dispositif est donc bien un dispositif transitoire, il sera revue dès que possible un nouveau directeur a été nommé à la tête du groupement, je pense que vous vous êtes au courant, je vous le partage si telle n'est pas le cas,

et et ministères seront mobilisés à ses côtés, évidemment, et nous continuerons à ce ces élus locaux, je n'ai pas d'août hein sur le directeur de Beauvais qui a été nommé par intérim sur le GHB Esso donc s'occupe déjà de BE de boeufs, de Beauvais et du GSPC, je n'ai pas de doute sur la volonté du directeur général de l'ARS, ce qui, une fois n'est pas coutume je suis obligé de le dire, simplement il faut leur donner des moyens exceptionnels pour pouvoir recruter et obliger à ce que ces médecins arrivent sur ce territoire parce qu'on est quand même à 50 kilomètres de Paris, c'est le le l'hôpital le plus proche de l'aéroport et l'autoroute A1, l'aéroport de Roissy, donc vous savez, c'est quand même un enjeu essentiel, surtout dans cette période Covid. Merci beaucoup, la parole est à monsieur Loïc Hervé pour la question orale numéro 1968 au ministre des solidarités et de la santé. Merci madame le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce matin, monsieur le ministre je veux évoquer la question de la grande précarité dans laquelle se trouvent les établissements médico-sociaux de la Haute-Savoie, alors que ces établissements : manque de personnel pour fonctionner de façon normale, les perspectives de recrutement sont inexistantes, résultat d'une situation tant conjoncturels et locales que structurelle, ce secteur souffrent d'un manque de reconnaissance et d'attractivité, d'autant plus qu'ils ne bénéficient pas du plan de revalorisation du Ségur de la santé ainsi des décisions drastiques et inhumaines, ont dû être prises contre la fermeture d'accueil temporaire et une prison ou alors une prise en charge plus courts, des occupants à la maison Notre-Dame de de l'Ordre de Malte à Sallanches, qui accueille des à des autistes, l'extension de 10 places inauguré en 2020 reste désespérément vides, faute de personnel suffisant malgré les opérations de formation réalisé avec les Greta, elle j'ai visité cette maison avec le député de la circonscription, Xavier Roseren et je peux vous assurer que le désarroi des familles est grand, que comptez-vous faire, Monsieur le Ministre. Merci monsieur le ministre. qu'elle s'explique en partie par la situation géographique de la Haute-Savoie, à proximité de la Suisse, et donc avec cette attractivité salariale qui séduit de nombreux professionnels du secteur, il est par ailleurs connu que les prix élevés en matière de logement en Haute-Savoie, je crois qu'il fallait dire pénalise également les installations, la nouvelle vague épidémique accentue encore ces tensions, les besoins de remplacements sont nombreux et bien donc accentuer la charge de travail de professionnels qui sont déjà éprouvée, la masse Notre-Dame de filet armes que vous avez cité connaît effectivement d'importantes difficultés cet établissement dans l'extension de 10 place a recueilli l'avis favorable de la commission consultative départementale de sécurité d'activité trouve ne trouve pas, pour l'instant de l'équipe nécessaire, c'est le point que vous souleviez alors en attendant l'ouverture effective le financement était reporté sur la création d'une équipe mobile autisme adulte. Intervenant depuis 2018 auprès d'aidants familiaux et professionnels, cette équipe incontournable sur le territoire, je crois, a été pérennisé lors du passage de l'organisme gestionnaire sous ses pommes alors l'ARS, oeuvre à réunir par ailleurs les conditions disponibilité de la ressource humaine avec la mobilisation de de différents leviers mutualisation des ressources avec les USMS, centre hospitalier l'HAD des services à à domicile, possibilité de passer des contrats de vacation de gré à gré avec des professionnels de santé libéraux, voire les faire participer au système et puis à moyen terme, il s'agira d'améliorer l'attractivité des métiers, vous le savez la mise bourguignon mène en la matière une action continue et déterminer le Ségur le plan métiers du grand âge et de l'autonomie ont permis d'importantes revalorisations salariales, le renforcement des formations mais aussi le lancement d'actions de communication sur les métiers du grand âge, avec d'ores et déjà des déclinaisons régionales pour faire connaître ces métiers essayer d'attirer 2 nouveaux candidats déclinaison qui se poursuit puisqu'une concertation est organisée en très différents acteurs impliqués sur le département de Haute-Savoie afin de définir ensemble une stratégie qui soit coordonné structuré et efficace. Merci. Si Monsieur Hervé, vous avez 54 secondes. Merci madame le président, monsieur le Ministre, j'entends votre réponse et le diagnostic, nous le partageons ainsi que les pistes de travail, le problème c'est que quand vous êtes confronté à à une maman seule de 80 ans, qui reprend à la maison, son fils autiste de 50 ans qui étaient habitués à vivre dans un dans un dans cette maison Notre-Dame de filières où il avait son cadre de vie habituel, ses habitudes et et que cette personne rentre rend revient à la maison et qu'elle est aux prise en charge par cette maman qui n'a plus les capacités d'énergie, de même, malgré sa générosité malgré son instinct maternel qui est indéniable, c'est un exemple humain dont je que je voulais que je voulais mettre en exergue ce matin pour vous dire vraiment quel est le désarroi de ces familles et il faut que pour la Haute-Savoie, à l'instar de ce que Amélie de Montchalin veut faire pour la fonction publique, on ait des réponses spécifiques les, les, les questions nationales ne répondront jamais à la typicité notre département merci. Merci, la parole est à monsieur Christian Billac pour la question orale 1841 au ministre des solidarités et de la santé. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues. La mise en place à janvier 2020 de l'avenant numéro 6 à la convention nationale des infirmiers libéraux avait pour objectif de garantir l'accès aux soins pour tous les patients de moderniser l'activité libérale et la simplification des actes infirmiers notamment en milieu rural et dans les territoires ruraux, les citoyens, on peut mesurer le rôle joué par les infirmiers libéraux dans cette période de crise de sanitaires non seulement sur le pas de la santé, mais aussi sur celui du vieil social et pourtant le Fatah qui ne tient pas compte de la réalité quotidienne dans la pratique de cette profession ainsi le dispositif du plafonnement journalier du montant facturé des anneaux métiers kilométrique porte préjudice à la profession, avec un abattement de 50 % à partir de 300 kilomètres dans demande de 5 % au-delà,

du Mountaga Tagada de la rémunération pour les infirmières décourage les plus jeunes de s'installer dans le milieu rural et on ainsi des déserts médicaux, c'est pourquoi monsieur le ministre, je vous demande de prendre des mesures urgentes pour revaloriser les prestations des infirmiers libéraux et en particulier sur ce problème des indemnités kilométriques et traduit réussir la reconnaissance de la profession. Bien que vous attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de revoir les dispositions de cet avenant, 6 à la convention nationale des infirmiers libéraux qui relatives notamment à la prise en charge des. Des indemnités kilométriques, considérant que celle-ci notamment ce ce dispositif de plafonnement journalier du montant facturé des indemnités pourraient être défavorables, en particulier dans les zones rurales et en particulier dans cette période de crise sanitaire a un Aamodt un abattement au tarifs de remboursement de ses indemnités est en effet déterminé au regard de la distance journalière facturé par l'infirmier, cette nouvelle disposition a pour objectif de limiter les difficultés qui existait effectivement précisé précédemment, ainsi que les uns du général, à ce titre, de laisser la possibilité pour de nombreuses affaires libéraux de de facturer ce qu'on appelle en étoile, c'est-à-dire sans mesurer à chaque fois, la distance à partir du du cabinet ce mode de calcul qui a été le fruit des négociations menées avec les représentants des infirmiers libéraux apportent donc en réalité une souplesse qui nous semble bienvenue et qui semble bienvenue à à tout le monde, c'est une disposition qui fait l'objet d'un suivi entre l'assurance maladie et les représentants des professionnels comme toutes les mesures conventionnelles d'ailleurs et pourra faire l'objet d'adaptation, le cas échéant par ailleurs souhaite souligner que des mesures ont été prises concernant l'accès aux soins qui est un des objectifs prioritaires du plan ma santé 2022, vous le savez l'avenant 6 permet à ce titre, d'améliorer la prise en charge et l'accès aux soins des patients en mobilisant plusieurs leviers: développement de la coordination pluri-professionnelles, l'investissement dans la prévention ou encore une meilleure connaissance des soins infirmiers, c'est la question des zones rurales que vous soulevez, enfin les mesures démographiques visant à un meilleur maillage territorial ont été renforcés pour favoriser l'exercice des infirmiers à ces endroits spécifiquement je peux citer par exemple l'aide forfaitaire à l'installation, qui s'élève à un montant de 27500 euros l'aide forfaitaire à la première installation qui, elle, de 37500 euros ou encore le contrat d'aide au maintien d'un montant de 3000 euros par an voilà nous prenons, je le crois, Monsieur le Sénateur, le mieux possible les spécificités des territoires.

et donc il ne gagne pas non plus de de rémunération quand et conduire leur voiture. Merci beaucoup, merci, je suspends juste quelques instants pendant que la ministre arrive, merci, merci Monsieur le mini.

La séance est reprise et je donne la parole à monsieur Didier Marie pour la question orale, numéro 2 1057 au ministre de l'Intérieur. Merci madame la présidente, madame la ministre à plusieurs reprises, notamment en décembre 2000 avril 2021 ainsi qu'au lendemain d'une rixe entre jeunes ayant causé la mort d'un d'entre eux, en juin 2021, les maires de la métropole de Rouen, de toutes sensibilités et moi-même vous alertons sur la montée de l'insécurité, les maires font tout ce qu'ils peuvent pour assurer la tranquillité publique, plus de policiers municipaux élargissement la vidéoprotection augmentation des actions de prévention mais ils ne peuvent se substituer à la police nationale, ces alertes sont restées sans réponse, la situation continue de se dégrader, augmentation du trafic des vols, des violences urbaines, des violences intrafamiliales exacerbée par le contexte sanitaire après ces alerte la préfecture a réalisé un important travail d'évaluation des besoins, confirmant la nécessité d'une augmentation du nombre de policiers en octobre dernier, le ministre de l'Intérieur finale a finalement annoncé l'arrivée prochaine, pardon, de 60 agents supplémentaires sur le territoire de Rouen Elbeuf et il s'est personnellement engagé à venir présenter le calendrier de leur déploiement depuis rien ce nombre, nous sommes déjà sous-évalué, mais il est au moins tant que ces promesses soient tenues de précédentes annonces du même type avait été faite en 2019 par le précédent ministre sans jamais avoir été honoré, nous sommes en janvier 2022 madame la Ministre quand ses effectifs arriveront-ils dans l'agglomération de Rouen Elbeuf merci. Merci, la parole est à Madame, Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, surtout, Monsieur le Sénateur, en matière de sécurité, vous avez raison, les attentes des Français sont fortes et sont légitimes et c'est pour cette raison que vous le savez le gouvernement comme la majorité parlementaire, on en fait une politique prioritaire en voulant mobiliser tous les leviers de la prévention à la répression, avec des moyens qui sont massifs concrets et mesurables et avec encore cette année une hausse de 1,5 milliard d'euros du budget du ministère de l'Intérieur, je veux dire que ce travail et doit se mener évidemment avec les élus locaux et que nous agissons pour renforcer l'efficacité des forces de l'ordre avec de nouveaux moyens avec des outils juridiques adaptés avec des policiers mieux formés, mieux équipés, cette transformation du numérique, elle se poursuit avec, par exemple, le prochain lancement de l'application ma sécurité Point FR qui permettra à chacun d'avoir accès aux forces de l'ordre plus facilement, notamment dans le cas du chantier de la plante en ligne, les premiers résultats sont là, même si évidemment, nul ne peut songer à nier la violence et les incivilités et d'ailleurs, plusieurs élus en sont les victimes, très Direct, mais vous avez raison, Monsieur le Sénateur, la question des effectifs, elle est centrale, même si la politique de sécurité ne saurait-ce et c'est pourquoi, conformément aux engagements pris, nous avons recruté au cours du quinquennat près de 10000 policiers et gendarmes supplémentaires une véritables réserves opérationnelles de la police nationale va par ailleurs se mettre en place toutes les circonscriptions de police auront bénéficié d'une hausse significative de leur effectif sur la durée du quinquennat mais nous devons aussi pouvoir agir pour qu'il soit davantage sur le terrain là où les Français aspirent à les voir, c'est la négociation menée sur les cycles horaires avec la substitution des policiers et des gendarmes, par du personnel administratif et à travers ce chantier qui est important de la réforme de la procédure pénale et demain, avec la création d'un corps de greffiers, de police, comme annoncé à Nice par le président de la République, ce mouvement va encore s'amplifier, notre objectif c'est un doublement d'ici 2030, de la présence des policiers et des gendarmes sur la voie publique pour mieux renforcer la sécurité du quotidien s'agissant de la circonscription de sécurité publique de Rouen je vous confirme, Monsieur le Sénateur qu'elle bénéficiera d'ici la fin du présent semestres d'un renfort de 60 policiers fin novembre 2021 7 circonscriptions de police s'appuie sur un effectif opérationnel de 597 gradés et gardiens, auxquels s'ajoutent 20 policiers dédié au quartier de reconquête républicaine, des hauts de Rouen 617 agents, ils n'étaient que 500 fin 2016 je vous remette. Merci, Madame le Ministre. Monsieur Marie, vous avez 42 secondes. Merci madame la présidente, madame la ministre, votre réponse reste générale, nous avons besoin aujourd'hui d'une date, et comme je vous le disais, la situation sur le terrain et tendue dans ma commune à Elbeuf, ce ne sont pas moins de 5 vols à main armée qui ont été commis par un individu dans des commerces locaux, le maire et ses commerçants ont écrit au ministre de l'intérieur pour demander une plus forte présence de la police nationale, j'espère que cette fois-ci qu'ils auront une réponse tout comme j'espère que les maires du territoire de la métropole obtiendront une réponse rapide et la présence du ministre qui viendra annoncer lui-même le calendrier, je vous remercie. Merci, la parole est à monsieur Christian Klinger pour la question orale numéro 1961 la ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants. Merci madame la présidente, madame la ministre, les conditions d'attribution au conjoint survivant de la demi-part fiscale propre aux anciens combattants, relève de l'article 195 du code général des impôts, modifié par la loi de finances pour 2020 depuis le 1er janvier 2021 les veuves ou veufs dans sa combattants bénéficie de l'attribution de la demi-part fiscale à compter de leur 74ème année si et seulement si l'ancien combattant est décédé entre 65 et 74 ans, si cette avancée a été apprécié sur le moment elle se révèlent insuffisantes à l'usage, si j'ose dire, aujourd'hui, la différence de traitement entre conjoints survivants selon l'âge du décès de l'ancien combattant piétine un principe essentiel qu'on appelle le principe d'égalité entre les générations du feu ce principe fondamental de notre défense nationale c'est conjoint survivant d'un ancien combattant mort avant d'avoir 65 ans subissent donc une double peine : perte de leur conjoint et privation d'un droit légitime, ils font les frais d'une carence d'évaluation et de conditions restrictives imposées par des politiques publiques et nous amener de leur préoccupation, ce sont près de 15 % des veuves ou veufs d'anciens combattants qui sont concernés, 100 seulement, me direz-vous mais pourquoi n'auraient-ils pas droit eux aussi à la reconnaissance de la nation pour les services que feu leur conjoint a rendu, madame la ministre, à l'heure où le nombre de nos anciens combattants et vivent en dessous du seuil de pauvreté, à l'heure où les futurs anciens combattants rentre du Mali où se battent au Sahel, pourriez-vous nous dire ce que vous comptez faire pour remédier à cette situation. Merci, la parole est à Madame, Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser ma collègue, la ministre Geneviève Darrieussecq et ne peut pas être présentes ce matin, elle m'a demandé de pouvoir vous répondre à ce que je fais bien volontiers, celle-ci a d'ailleurs récemment clôturé le congrès de la fédération qui est à l'origine de l'enquête que vous évoquez, qui a veillé à entretenir depuis 2017 avec l'ensemble des associations d'anciens combattants des échanges nourris et fructueux, je veux d'abord bien sûr penser aux veufs et aux veuves de guerre aux invalides de guerre qui ont consenti par la perte de leur conjoint, l'ultime sacrifice et auquel nous devons évidemment une reconnaissance exemplaire et sans faille, c'est pourquoi d'ailleurs, il bénéficie d'une pension militaire pour pourvoir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants qui sont à leurs pupilles de la nation, il bénéficie aussi d'une demi-part fiscale sans condition d'âge pour eux comme pour le conjoint décédé au combat, par ailleurs, le ministère des Armées porté en 2000 19 et en 2020, des mesures favorables pour ces femmes pour ces veuves, notamment celles qui ont apporté des soins constants à leur conjoint invalide dans des conditions particulières, en 2022, c'est une augmentation exceptionnelle du point PMU de 14,70 à 15 0 5 euros qui a été décidée par le gouvernement, elle aura un effet visible et immédiat sur le niveau de vie des veuves et c'est là une mesure de justice pour celle ou pour ce d'ailleurs dont le conjoint n'a pas été blessée mais a obtenu la carte du combattant, la priorité a été pour nous d'augmenter, de maintenir les moyens de soutenir les plus fragiles, ces veuves qui généralement ne sont pas imposables doit faire face aux frais de la vie courante, parfois sur leur dépendance et, là, le budget de l'action sociale qui est essentielle, en complément de l'action résolue du gouvernement pour les petites retraites, je pense à l'augmentation de 100 euros par mois du minimum vieillesse, notamment en 2021, de nouveau, ce budget a été consommée, grâce à la mobilisation des services de proximité voici quelques priorités qui sont portées par le ministère délégué chargé de la mémoire et des anciens combattants, depuis 2017, à savoir d'une part la reconnaissance pour celles qui ont pris qui, pardon, qui par leur conjoint, hé bien ont consenti à cet ultime sacrifice et d'autre part par l'accompagnement des plus fragiles et qui est absolument essentiel, je vous remercie. Merci Monsieur Clean, vous avez 23 secondes. simplement pour vous dire ça représente vraiment une goutte d'eau hein sur le budget de l'État, on a dépensé des milliards ces derniers mois, on pourrait aussi penser à assez veuve et ses veufs, je rappelle quand même que la retraite d'ancien combattant, qui est une expression de la reconnaissance de la nation représente 782 euros par an. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Patrice Joly pour l'action orale, numéro 2000 49 ans, ministre des solidarités et de la santé. Merci madame la présidente, madame la Ministre, mes chers collègues, depuis le 1er janvier 2022 le forfait Passion, urgence entre en vigueur, il s'agit d'un forfait de 19 euros 61 facture à toute personne qui se rend aux urgences d'un hôpital pour soins non suivies d'une hospitalisation dans les idées, médicaux, il y a là une double peine pour les habitants, la première est liée à la possibilité pour ces habitants des territoires ruraux d'accéder à la médecine de ville et cela n'est pas près de changer, puisque le nombre de médecins qui pourraient partir à la retraite dans les 10 années qui viennent, atteint dans certains départements, des taux très élevés ainsi dans la Nièvre, les 2 tiers d'entre eux ont plus de 55 ans, répondre à répondre aux besoins des Nivernais alors qu'entre 2010 à 2017 le nombre de médecins avaient déjà diminué de 27 %, aujourd'hui il y a moins de 7 médecins généralistes pour 10000 habitants, pour 10000 habitants dans la Nièvre, sachant qu'une part importante d'entre eux exercent dans l'agglomération de Nevers à cette pénurie de médecins généralistes, il faut ajouter la disparition des gardes le soir et le week-end, le refus des quelques médecins restant à prendre de nouveaux patients faute de temps, les urgences peuvent donc souvent être unique recours proposer à la population pour se soigner, un autre phénomène encore plus inquiétant découle de ce forfait, l'action des inégalités sociales d'accès aux soins en effet les personnes les plus précaires au tarde malheureusement leurs soins faute de ne pouvoir accéder avancer les frais et se retrouvent conduit aux urgences dans un état très critique alors que cela aurait pu être évité aussi devant de telles inégalités territoriales et sociales d'accès aux soins et par l'incidence d'espérance de vie je vous demande, je demande au gouvernement, comme l'a fait, l'association des maires ruraux que les patients vivants d'une part dans les déserts médicaux et notamment issus du monde rural, et d'autre part, privée de médecins soient ajoutés à la liste des personnes exonérées intégralement de ce forfait, je vous remercie. Si la parole est à Madame, Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Si madame la présidente, monsieur le sénateur, je représente le ministre de la Santé et des solidarités Olivier Véran, il m'a chargé de vous répondre de sa part, vous appelez l'attention du gouvernement sur les conséquences de la mise en place du forfait Passion, urgence, notamment pour les personnes qui n'auraient pas accès à un médecin traitant, faute d'une densité suffisante de professionnels de santé, je vous dire d'abord que vous savez que le gouvernement est particulièrement concernés et sensibles à la nécessité de pouvoir garantir un véritable accès aux soins et ce sur l'ensemble du territoire, je veux rappeler d'ailleurs qu'une participation était déjà acquittés précédemment par les passions lors de leur passage aux urgences, il a mise en place du forfait Passion, urgence n'augmente pas les restes à charge mais elle simplifier les modalités de calcul de la participation à la forfait de 6 ans le montant de cette participation forfaitaire a été calibrée de manière à pouvoir maintenir le niveau moyen de participation à l'identique et permet notamment une meilleure protection des usagers nécessitant des soins complexes dont la participation pouvait avant d'atteindre un montant de 60 euros en moyenne, l'accès est toujours possible pour les patients, même si, bien sûr, ils n'ont pas leur carte vitale ou qui n'ont pas leur pièce d'identité par ailleurs ce forfait pris en charge par les complémentaires santé, la question des restes à charge les donc davantage liée à l'accès des assurés à une couverture complémentaire, seuls 4 % des assurés ne dispose pas d'une telle couverture et le gouvernement est pleinement engagée pour faciliter le recours à cette couverture, enfin, le gouvernement a voulu que la loi de financement de la Sécurité sociale de 2022 permettent l'attribution automatique ou simplifier de la complémentaire santé solidaire aux bénéficiaires de Revenu de Solidarité Active ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, je vous remercie. Merci monsieur Joly, vous avez 13 secondes. de santé faute de moyens, les soins seront donc repoussé jusqu'à pour ces personnes-là aggravation et donc jusqu'à l'hospitalisation, il est inacceptable que la santé de là aujourd'hui un luxe. Par ce forfait, cher collègue, la parole est à monsieur le président, Guillaume Gontard pour la question orale, numéro 2 1060 transmise à la ministre de la transition écologique. Oui merci madame la présidente, madame la ministre, pour conduire le chantier de la rénovation thermique des logements, le gouvernement mise sur le dispositif ma prime si les demandes sont nombreuses : 617000 l'an dernier et les besoins bien réelle, force est de constater que cette aide n'a pas les moyens de ses ambitions, d'abord elle ne concerne que très peu de rénovation globale on sait pourtant que c'est l'essentiel et que c'est des rénovations qui sont bien plus vite efficace en matière d'économie d'énergie, ensuite, malgré une hausse des effectifs de l'Anah, les délais de versement des primes sont beaucoup trop longs, ainsi, seuls 294000 primes ont été versées l'an dernier, soit un peu moins de la moitié alors que vous avez fixé le délai d'instruction des dossiers à 2 mois le délai moyen est aujourd'hui de 5 mois et 8 et 8 % des dossiers prennent même plus d'un an, les bénéficiaires sont alors obligés d'avancer plusieurs milliers d'euros pour leurs travaux, ils peuvent se retrouver en grande difficulté financière beaucoup de dossiers sont bloqués ou pire sont jugées irrecevables en raison d'erreurs involontaires dans les documents 36 transmis par exemple une erreur de quelques jours sur la date du devis ou un défaut de renouvellement des certification RGE par les professionnels, la rigidité des critères prévus pour lutter contre la fraude, a des conséquences financières catastrophiques et décourage de nombreux bénéficiaires, souvent les plus démunis à s'engager dans la réalisation de travaux de rénovation alors que le gouvernement a créé un droit à l'erreur en 2018 pour aider les entreprises, pourquoi ne pas appliquer les mêmes règles aux citoyens de bonne foi, de nombreux citoyens témoigne d'importantes difficultés à joindre la la Lana, notamment en raison du recours à la société d'aucun poste, en effet, les dossiers sont traités par cette entreprise sans communication interne des 2 des demandeurs font souvent face à un service déshumanisé et un suivi erratique alors Madame la Ministre, comment le gouvernement compte assurer un traitement à la fois humain et efficace des dossiers et un versement rapide des aides à nos concitoyens, Merci, la parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci, bonjour madame la la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Gontard, je crois que personne ne peut. Ne peut. Revenir sur le fait que cette prime rénove, elle rencontre un succès indéniable, et pour cause : nous avons en 2021 plus de 760000 dossiers qui ont été déposés 660000 ont été engagés pour un montant de plus de 2 milliards d'euros, c'est quelque chose de considérable non seulement au niveau budgétaire, au niveau de cet engagement financier de l'État, aux côtés de ces ménages mais aussi dans le volume de dossiers déposés, c'est dire les attentes et et si elle rencontre vraiment un un succès extrêmement fort évidemment quelques dossiers peuvent poser parfois problème pour autant dans leur grande majorité, une fois la validation de l'reçu les projets, les ménages réalisent leurs travaux envoie la facture sur ces ces travaux finis et reçoivent ma prime rénove, il est évidemment normal que toutes les aides, engagées en 2021 n'est pas encore été versée, mais ce sont tout de même à ce jour 370000 ménages ayant fini leurs travaux qui ont été payés en en 2021 alors à date, nous avons plus de 99 % des dossiers déposés complet qui sont traités dans les 15 jours je vous rejoins sur la nécessité de regarder les dossiers qui peuvent être plus plus difficile et plus complexe, ce que nous faisons et ces dossiers nécessitant des échanges s'ils ne sont pas complets ou présentent des erreurs sont traités donc après une décision rendue en moyenne en en 30 jours ouvrés, nous avons donc intégrer ce temps de retour des ménages sur leur sollicitation et cela concerne aujourd'hui moins de la moitié des des dossiers à l'engagement, trouvé ce dispositif de la plus grande réactivité sur des dossiers qui seraient incomplets ou contenant des erreurs avec un délai moyen de paiement qui est 18 jours en prenant en compte les contrôles sur place, des contrôles qui sont évidemment indispensables pour lutter contre d'éventuelles fraudes par ailleurs, les enquêtes de satisfaction sont sans conteste conteste pardon je crois puisque nous avons 89 % des bénéficiaires qui sont déclarés satisfaits de ma prime rénove avec 84 % satisfaits du respect des délais annoncés, j'entends donc vos points d'alerte sur sa maison, point de détail mais je crois que globalement tout le monde est félicite de ce dispositif. Merci monsieur le président Gontard vous savez 9 secondes. Oui merci madame la Ministre, non, moi je voulais juste vous alerter effectivement sur des des cas particulièrement graves avec des personnes à très faibles revenus et qui se trouvent dans des situations particulièrement compliqué, je pense qu'il faut y porter quand même attention, même si, effectivement, c'est pas la majorité. Merci, la parole est à Madame Christine Herzog pour l'action numéro 2016 à la Ministre délégué chargé du logement, la présidente. Madame la ministre, mes chers collègues, de nombreuses ancienne région minière et industrielle comme la Moselle possèdent des logements anciennement destiné aux ouvriers et appelé Familistère ces logements haut depuis le depuis le XIXe siècle, changer de propriétaire passant de propriétés des usines à celle des ouvriers eux-mêmes qui ont alors pu acquérir leur propre logement, ces habitations sont à la rentrée, dans la catégorie des résidences privées mais cette opportunité est rapidement devenue un cadeau empoisonné ses nombreux propriétaires ne constitue pas une classe sociale supérieure et sont de plus souvent ouvriers parfois retraités disposant de très faibles revenus, ses 13 de 13 de cette très ancienne construction devenu au fil des années des passoires thermiques qui ont un coût très important pour les familles qui les habite, considérés comme des résidences privées les communes ne peuvent pas aider les occupants de la réparation de ces habitations puisqu'elles ne sont pas éligibles ni en financement attribués aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, dits QPV, ni à l'aide massive de l'Agence nationale de rénovation urbaine comme c'est le cas pour les bailleurs sociaux des habitants à loyer modéré, un autre problème se pose celui de la mixité sociale, la loi SRU impose un minimum de 20 % de logements sociaux aux communes, or ces anciens familistère qui sont désormais des résidences privées ne correspondent pas aux critères, bien que les populations qui habitent ne soient pas financièrement aussi, pourriez-vous nous indiquer, madame la ministre, si dans le cadre de la nouvelle contractualisation de la géographie prioritaire de la politique de la ville, allant de 2014 à 2024 abondé de 5 milliards d'euros, ces quartiers au statut très particulier, pourront en bénéficier à être pris et être pris dans les quotas sociaux des communes comme la loi SRU n'impose. La parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs Madame la la sénatrice Herzog cette réhabilitation des anciens logements ouvriers situés dans dans les anciens Familistère que vous mentionnez notamment Anne il vend Jean Moget en Moselle et représente effectivement un enjeu que vous avez réellement raison de souligner parce qu'effectivement, dans le cadre de l'ANRU du programme de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, ils ne peuvent pas bénéficier de ces aides, à savoir qu'ils ne sont pas identifiés dans la liste des 480 quartiers prioritaires de la politique de la ville, éligibles au nouveau programme de de renouvellement urbain, qui a été institué par la loi du 21 février 2014 et il semble difficile aujourd'hui de revoir ce ciblage de ce programme, à ce stade, en revanche, ces logements sont bel et bien éligible aux aides des dispositifs de l'Lana de l'Agence nationale de l'habitat dont la vocation est justement de traiter ces situations, la rénovation de l'habitat privé, c'est une priorité de ce gouvernement, vous le savez, nous avons agi fortement dans le cadre de de dispositifs existants, tout en améliorant les financements à destination des plus modestes, ma prime rénove pour les travaux sainte à ma prime rénove sérénité pour des travaux plus globaux et lourd et complexe qui touche très directement, parfois des logements indignes et puis également au plan d'initiative copropriété qui apportent des financements renforcés pour diminuer le reste à charge dans le cas de copropriété réhabiliter les les immeubles dégradés avec plus de 500 millions d'euros qui ont été versées dans ce cadre, ce sont presque 100000 logements qui ont pu être réhabilités les opérations programmées de l'habitat, porté par l'Anaes, sont également un outil utile dans ce cadre d'ailleurs la communauté d'agglomération du Val de Fensch envisage précisément dit dit recouvre d'y recourir et puis concernant la la prise en compte des logements concernés au titre de la loi de solidarité de renouvellement urbain, la SRU, elle est essentiellement assis sur le conventionnement APL qui garantit un statut locatif social Claire alors une solution pourrait être l'acquisition totale ou partielle du Patrimoine par un bailleur social ça permettra effectivement de répondre à ce triple objectif de la rénovation des logements par le bailleur du développement d'une offre abordable et de leur comptabilisation à l'inventaire SRU ce type de montage, il pourrait d'ailleurs utilement s'appliquer aux patrimoines des cités ouvrières, dès dès lors que les propriétaires ou les communes souhaitent vendre ces logements, je vous remercie. Merci, la parole est à monsieur Hervé Maurey pour la question orale, numéro 2022 à la ministre de la transition écologique. Madame la présidente, madame la Ministre, cela fait maintenant 5 ans que le Sénat alerte régulièrement le gouvernement sur la dégradation inquiétante de nos infrastructures, de rapports sénatoriaux ont été publiés, l'un sur l'état des routes en 2017, l'autre sur l'état des ponts en 2019 malgré ces mises en garde l'état des infrastructures continue à se dégrader, comme en témoigne l'édition 2021, du rapport de l'Observatoire national des routes cet entretien et pourtant un enjeu important en terme de sécurité routière déjà puisque le mauvais état des infrastructures est impliqué dans un quart des accidents de la route et c'est également un enjeu en termes financiers, puisque lorsqu'on investit pas un Euro aujourd'hui, c'est un terme 10 euros, qu'il faut investir dans l'infrastructure, si quelques efforts budgétaires ont été consentis, nous sommes très loin du compte, puisqu'il manque 100 millions d'euros en 2022 par rapport aux besoins estimés par l'État lui-même sur le réseau routier non concédé quant aux communes et aux intercommunalités qui ont la responsabilité de 2 tiers du réseau routier français, elles sont que faiblement et parfois même pas du tout aidé par l'État dans le cas du plan de relance 40 millions d'euros sont prévus pour les aider à entretenir les ponts 40 millions on est très loin des 130 millions par an que nous jugeons nécessaire dans notre rapport, ma question est donc très simple Madame la Ministre, pourquoi, malgré les mises en garde du Sénat à voir ainsi se laisser se dégrader l'état de nos infrastructures, infrastructures, pardon, au risque de mettre en danger la sécurité de nos concitoyens. Merci, la parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Maurey si j'ignorais votre implication sur ces questions et de longue date, je je serais beau beaucoup plus directe : je sais votre souci et je vous réponds également en tant qu'ancienne, rapporteur de la loi d'orientation des mobilités, sur le volet précisément du financement des infrastructures avec une priorité dont vous avez convenu, je crois, dans cette loi d'orientation des mobilités une priorité à la rénovation de l'existant, qui avait souffert d'un large sous-investissement pendant des décennies, et vous le savez, et cette priorité, elle s'est traduite dans les chiffres, puisque les les crédits dédiés, assez, assez, rénovation de l'existant, on consomme ont considérablement augmenté, tout d'abord, alors s'agissant du réseau routier national, vous le savez, nous avons rendu public dès 2018 les données dans un souci de transparence pour que chacun effectivement aient accès à cette photographie de l'existant. Qui était effectivement extrêmement inquiétant, avec également des audits indépendants qui ont été menées sur l'ensemble du Patrimoine existant pour quantifier ses besoins en terme de d'investissement, travaux qui ont été publiés et qui ont guidé les choix du gouvernement et du du le comité d'orientation des infrastructures auquel vous avez largement apporté votre concours, dans ce cadre, le gouvernement a décidé vraiment d'accorder cette priorité à l'entretien du réseau existant, avec une priorité aux ouvrages d'art, un effort financier sans précédent que vous connaissez puisque l'entretien du réseau routier non concédé est passé de 708 millions d'euros en 2017 à 850 nous avons donc vraiment un effort très conséquent qui s'ajoutent aux 40 millions supplémentaires mis en oeuvre dans le cadre du plan de relance de l'économie 2000 22 et grâce auquel des chantiers pluri-de réparation de cet ouvrage importants ont pu être sit-in flic hâtivement accéléré comme par exemple le le viaduc d'autres villes ou sur le l'autoroute A31 en Meurthe-et-Moselle, avec donc l'ensemble des infrastructures du réseau national qui est sous surveillance permanente tous les ponts du réseau routier national sont désormais sous sous surveillance avec des visites annuelles et des inspections, il n'y a pas de situation d'urgence avérée, mais une vigilance accrue aujourd'hui et, et, s'agissant des des réseaux routiers, vous savez que nous y sommes. Particulièrement vigilants, madame la ministre, je vais vous rappeler à l'ordre sur le temps parce que 10 secondes à chaque seconde, voire 15 c'est juste pas possible monsieur Morin, vous avez 24 secondes. Bien en en 24 secondes je, je dirais même la même liste que je ne nie pas et je l'ai dit qu'il y a eu des efforts de faits, je dis simplement qu'ils sont très insuffisants, puisque au regard des chiffres fixés par l'État lui-même, il manque 100 millions pour l'entretien du réseau routier national et que, en ce qui concerne les ponts, on avait mis, vous aviez mis 60 millions en loi de finances 2021, c'est passé à 40 en loi de finances 2022, et il faudrait 130 par an, donc voyez qu'on est très loin du compte, donc, pour résumer, avant que Madame la Présidente, ne me rappelle à l'ordre et des efforts ont été faits mais peut largement mieux faire. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Pierre-Jean Vergne Solenne pour la question orale, numéro 2 1029 à la ministre de la transition écologique. Madame la présidente, madame la ministre ma question porte sur l'éolien ce plus particulièrement sur les nuisances nocturnes qui sont liées à l'éclairage en haut des mâts la nuit qui sont pénibles pour les riverains qui sont déstabilisants des fois d'ailleurs pour ceux qui conduisent bien certains endroits sur le territoire ou en tout cas dans l'aine ou à certains moment, on voit plus, on ces éclairages, ils sont liés à des questions de sécurité par rapport au par rapport à l'aviation, il y a des expérimentations qui ont été lancées il y a maintenant maintenant quelques temps qui permettrait de limiter ses ces nuisances soit un éclairage aux extrémités des parcs, soit des éclairages qui se déclencheraient à l'arrivée des avions avec des détecteurs qui serait et dans les avions et dans le parc éolien et troisièmement sur une autre forme d'éclairage qui partiraient plus vers le ciel et moins moins de manière latérale, je voulais savoir, Madame la Ministre, où en étaient ses expérimentations et est-ce qu'une gêne la généralisation est prévue, merci de votre réponse. Merci Madame Bérangère Abba, vous avez la parole. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le, le sénateur Vert alors effectivement ce balisage des parcs éoliens, il est obligatoire, vous le savez, pour des raisons évidentes de sécurité, des aéronefs, mais nous, nous devons trouver le bon équilibre entre cette nécessité de sécuriser ses installations et la sécurité aérienne avec l'acceptabilité locale des des projets éoliens et je vous épargne les impacts également en termes de de biodiversité de la pollution lumineuse des émissions lumineuses notamment à éclats qui ne constitue pas une nuisance excessif pour les, pour les riverains des expérimentations qui ont été réalisés sur des parcs en service sous l'égide d'un groupe de travail réunissant des risques de représentants professionnels de la filière éolienne, les services de l'aviation civile et le ministère des Armées et des évaluations en vol réalisé au 1er semestre 2021 notamment en Ardèche sur le parc de Freycinet, qui ont permis de valider l'acceptabilité de feu dont les faisceaux ont été modifiés pour émettre moins d'intensité lumineuse en direction du sol et des des riverains avec d'autres évaluations qui sont menées sur le parc de choquer en Vendée par exemple ou de planer, en Ardèche, qui étudie les possibilités, diminution de la fréquence des éclats lumineux, combiné à la réduction de l'intensité les conclusions de ces campagnes de vol, elle devrait être connu au au 1er semestre au 1er trimestres pardon 2022, donc très prochainement pour savoir si les configurations testées ont été jugées acceptables ou si de nouvelles évolutions sont possibles et nécessaires, alors les les évaluations en cours d'organisation sur le site de sources de Loire en Ardèche pour étudier les possibilités de déclencher les feux de balisage nocturne uniquement au passage des aéronefs, ce qui diminuerait fortement également les les impacts sur les riverains ces évaluations seront menées au 1er semestre 2022, alors nous sommes bien conscients un Inde de ce problème que vous soulevez pleinement impliqués dans ces expérimentations avec des nouveaux types de de feu à Faissault qui seront prochainement autorisés à l'occasion d'une mise à jour de la réglementation relative au balisage des obstacles à la navigation aérienne, et puis des exploitants de parcs éoliens qui pourront toujours commencé le le déploiement de ces balises avec un déclenchement donc du balisage uniquement au passage d'un aéronef qui pourrait progressivement être généralisée à partir du second semestre 2022,

donc on a bien compris que les choses avancent et évidemment on vous invite à ce que les choses puissent rapidement se généraliser sur les nouveaux projets, mais également sur toutes les éoliennes qui ont été montées de depuis quelques années. Merci, la parole est à monsieur le président, Jean-François Rapin pour la question orale, numéro 2 1052 à la ministre de la transition écologique. Madame la présidente, madame la ministre ma question porte sur les communes concernées par le recul du trait de côte, sous l'autorité des préfets de département une délibération des conseils municipaux a été sollicité dans un délai de seulement quelques semaines pour permettre la publication d'un décret qui fixera la liste des communes dont l'action doit être adaptée au recul du trait de côte, de nombreux maires refusent de délibéré sans avoir pleinement connaissance des critères utilisés et des conséquences qu'importe ce décret, en effet, ces élus ne dispose d'aucune information sur les études qui ont été conduites par le ministère ni de précisions sur les conséquences du classement, lesquels dépendant d'ordonnances non publiés, malgré les réunions organisées en urgence par l'État sur les territoires, qu'en sera-t-il de la décote administré de la valeur des biens exposés au recul du trait de côte, quelles seront les conditions pour mener les relocalisations spatiale à l'échelle des communes, ces informations préalables sont indispensables pour la validité des délibérations et pour l'exercice de la démocratie locale, par ailleurs, la loi prévoit la possibilité pour les collectivités concernées de conclure une convention avec l'État afin de préciser les moyens techniques et financiers mobilisés pour accompagner les actions d'adaptation au recul du trait de côte, la note diffusée par les services ministériels prévoient que le dispositif de financement fera l'objet d'une communication ultérieure, à ce jour, la loi de finances pour 2022 n'a apporté, n'a pas apporté les réponses attendues dans ces conditions, il est urgent de prévoir un report de la consultation, sollicité par les préfets, il ne s'agit en aucune manière de nier les enjeux et la nécessaire adaptation de nos territoires mais en portant la parole des maires et des élus du littoral, je vous demande formellement de leur faire parvenir les études scientifiques permettant de justifier leur inscription sur cette liste et les réponses attendues bien sûr aussi sur le financement Madame. Merci, la parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur a pas cette anticipation l'érosion littorale, elle est, elle est essentielle, tout le monde partage aujourd'hui cette cette pour ne pas aggraver la Villeneuve la vulnérabilité des territoires et pour préserver au maximum le nombre de biens qui pourraient être exposées cette anticipation elle repose d'abord sur l'identification des communes les plus. Posez vous l'avez dit, avec des réunions d'informations qui ont été réalisées par les préfets au niveau local pour expliciter les critères d'élaboration de la liste et accompagner les les collectivités évidemment quand de besoin il faut ressusciter les préfets pour des informations supplémentaires, mais je vais être plus complète, compte tenu du contexte particulier, notamment de la situation sanitaire, le délai de retour des consultations qui était fixée au 24 janvier va être adapté pour laisser du temps aux communes pour réunir leurs conseils municipaux et pouvoir en débattre avec une anticipation qui repose également sur l'élaboration d'une cartographie locale d'Exposition au recul du trait de côte, une réforme nécessaire également de l'information des acquéreurs locataires cette cartographie, c'est bien la seule obligation qui s'impose aux collectivités listés et qui peut être vraiment dans ce dans certains cas un 1er pas vers une prise de conscience de de cette Exposition majeure à ce à ce risque, le gouvernement a été donc habilité à prendre des dispositions complémentaires par voie d'ordonnance ces écritures, elles sont en cours d'élaboration avec principalement des points sur la création d'un nouveau régime de bail réel immobilier des méthodes méthodes d'évaluation des biens et également des dérogations ponctuelles à la loi littoral, ces mesures, elles visent vraiment à faciliter les démarches de recomposition territoriale, elles viendront uniquement préciser les contours de ces outils dans l'utilisation restera à la discrétion des collectivités territoriales, elle ne crée pas en aucun cas de nouvelles obligations cette délibération des communes, elle est bien circonscrite à la reconnaissance de la particulière Vullnet vulnérabilité de leur territoire, ainsi que des activités bien qui sont exposés et non sur leur engagement à recomposer le le territoire c'est donc vraiment un outil de pédagogie et de de d'entraînement de prise de conscience et de projection dans ce que pourraient être ces atteintes avec au plan financier, l'État, qui s'est engagé à cofinancer les cartographies jusqu'à 80 % il est donc possible de mobiliser ses projets de manière partenariale. C'est monsieur le président, vous avez 18 secondes. Merci madame la présidente, madame la Ministre, hein, j'ai bien entendu que le délai était reporté, merci donc merci au 1er ministre à qui j'avais écrit récemment, deuxièmement, hein, il ne faut pas dire qu'il y a eu des réunions de concertation préalable à l'élaboration de ces listes, ça n'est pas vrai, des réunions sont venus après parce que les maires se sont affolés, troisièmement, sur le financement, il est bien discret, Madame la Ministre et quatrièmement, il est bien discret, effectivement, il y a rien au PLF et quatrièmement, je pense que les ordonnances aurait dû venir avant, on aurait dû connaître les ordonnances avant déterminant. Consultation merci madame, merci, la parole est à Madame Florence risquons comptable pour la question orale numéro 1903 la ministre de la transition écologique. soutien aux centrales villageoise, l'arrêté du 6 octobre 2021 fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations photovoltaïques inférieures à 500 kilowatts cet arrêté interdit de cumuler le rachat de l'électricité produite au tarif garanti et une subvention par une collectivité locale, c'est l'article 13 il met par la même en difficulté de nombreuses initiatives locales, notamment les centrales villageoises vertueuse pour la transition énergétique, nous nous avons, dans mon département, de la plusieurs expériences concrètes et positives, je partage le souci de veiller au respect des traités européens, toutefois, à l'heure du Green deal, les autorités européennes doivent prendre en compte l'apport citoyen que ces initiatives manifeste pour la transition énergétique ces initiatives citoyennes et locales ne dispose que d'un investissement initial associatif parfois complété d'un prêt sur 15 ans et doivent s'appuyer sur un important travail réalisé par des bénévoles, le soutien des collectivités permet d'engager les frais de raccordement au réseau d'assurer la viabilité des projets, y compris vis-à-vis des organismes prêteurs ces installations de taille réduite ne sont en aucun cas en concurrence réelle avec les grands opérateurs mieux, elle permet de faire émerger des projets de production d'énergie renouvelable, sur l'ensemble du territoire et elles ont besoin pour être économiquement viable d'un soutien d'amorçage limité à quelques exercices soit un seuil pertinent, Madame la Ministre, comment entendez-vous corriger les effets désastreux de cet arrêté afin de soutenir ces initiatives initiatives vertueuse, le plus souvent associatives, citoyennes et locales. merci, merci pour votre question parce que je partage tout à fait votre ambition est vraiment une certitude, celle que ses projets d'énergie quand ils sont citoyens ils impliquent largement la population et c'est comme ceci également que nous pourrons parvenir à cette transition écologique qu'il appelle une montée en puissance des des ENR et qui ne sont jamais aussi apprécié et accepter que compte cette énergie est partagé et et ses projets co-construits avec donc dans ses objectifs climatiques que nous partageons, plusieurs dispositifs de soutien financier aux installations d'énergies renouvelables, des dispositifs qui constituent des aides d'État et comme vous l'avez dit, ces aides, elles doivent être validées par la Commission européenne avec des décisions européennes de validation qui prévoient généralement une interdiction de cumul avec d'autres aides, notamment de régimes locaux, régionaux, nationaux ou de l'Union européenne cette condition, elle vise à garantir que la rémunération du producteur d'électricité restent raisonnables, ce qui est ce qui est une exigence du du droit européen, mais aussi du droit français, c'est un tiers de diction, de cumul, elle n'est donc pas une nouveauté, hein, de l'arrêté tarifaire d'octobre 2021, elle existait déjà et et elle doit s'interpréter vraiment dans le sens de l'interdiction de cumuler des aides à l'installation, les éventuels soutien relatifs à des aspects du projet qui ne sont pas couverts par l'arrêté tarifaire reste possible, par exemple, cumulé le tarif d'achat d'électricité avec des aides pour la préparation des terrains ou des structures qui pourraient être délivrés en l'absence de projets d'énergies renouvelables, cela inclut par exemple des aides à la rénovation de la toiture pour permettre l'accueil de panneaux photovoltaïques le cumul avec une aide pour certains coûts surtout pardon surcoût également en terme de raccordements électriques par rapport au projet classique est également envisageable et puis étant donné que l'arrêté du 6 octobre 21 ne comporte pas d'aide spécifique pour le projet citoyen, les collectivités locales peuvent verser des aides supplémentaires pour compenser les surcoûts liés au caractère citoyen des projets, notamment sur la mobilisation de la communication, la concertation, et même pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour leur permettre d'être économiquement viable en comparaison à des projets plus classique, nous avons donc un panel d'aide qui peuvent être mobilisés vraiment pour maintenir cette dynamique de projet citoyen, avec également des bonus dans la notation dans la notation des appels de. Merci à un ami faudra réajuster vos fiches à 15 secondes en moins madame quant vous avez 19 secondes. Merci madame la ministre, je j'ai bien entendu votre réponse cède à l'installation sont essentiels, souvent pour la viabilité de ces, de ces initiatives et aux assises de l'énergie citoyenne, madame la ministre de la transition écologique un ticket vouloir 1000 initiatives citoyenne, je constate sur le terrain que ces dispositions coupe les pattes à ceux qui démarre et c'est quand même très regrettable pour atteindre ces objectifs. Merci, la parole est à Monsieur, Cédric Vial pour la question ranimeront 1963 au ministre de l'Économie, des finances et de la relance. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, vous n'êtes pas sans ignorer que la Compagnie des Alpes est en train de développer une nouvelle stratégie qui n'est pas sans conséquences pour l'économie de la montagne, en effet, les récentes initiatives prises par la Compagnie des Alpes, et notamment la politique de développement de la chaîne de valeur dans les activités de montagne marque une évolution radicale au regard de la mission d'origine qui lui a été confiée par l'État en matière d'aménagement du territoire, cette diversification de l'activité de la Compagnie des Alpes, avec par exemple le rachat d'une importante école de ski ou encore l'affrètement de trains privés pour transporter les voyageurs qui auront acheté une de séjour pas caché par la CDA a des répercussions importantes sur l'ensemble des professionnels locaux de la montagne, pourtant la raison d'être de la Compagnie des Alpes, dont l'État est encore actionnaire à 40 % via la Caisse des dépôts et consignations était initialement de contribuer à l'aménagement et au développement des territoires de montagne et de l'ensemble de leur écosystème. Dans ce contexte, il est légitime de s'interroger sur l'évolution volontaire de ces missions ou le développement de l'autonomisation de cette filiale de la Caisse des dépôts et consignations, dont l'objectif est d'être et je site entièrement dédié au service de l'intérêt général, avec un objectif unique : faire grandir la France. Aussi je souhaiterais savoir si cette nouvelle stratégie a été validée par l'État et le cas échéant, quelle directive comptez-vous prendre pour encadrer cette diversification des activités de la Compagnie des Alpes, en veillant à ne pas gêner les acteurs locaux traditionnels de ce secteur, comment pouvez-vous également rassurer les élus et les acteurs économiques de la montagne sur le fait que les retombées économiques dont bénéficie la Compagnie des Alpes, en exploitant parmi les plus grands domaines, ce qu'il y a français et en maintenant mais maintenant en se positionnant sur ses activités concurrentielles avec des acteurs locaux continuent à bénéficier à l'objectif initial d'aménagement des territoires de montagne fixé par l'État à à cette compagnie, je vous remercie. Merci beaucoup, madame la présidente, mesdames et messieurs les les sénateurs et sénatrices et monsieur le sénateur, Cédric Vial, je crois que la la période que nous venons de traverser cette période de crise pandémique et de ses conséquences, a bien montré une chose dans le secteur du tourisme, c'est que le tourisme, c'est un ensemble d'acteurs qui, chacun, sont les maillons d'une chaîne, et si un des maillons vient à céder, c'est l'ensemble de la chaîne, qui peut également céder et donc j'évoque cela parce que c'est vrai aussi pour l'économie de la montagne et c'est pourquoi il y a, il est capital que chacun de ces acteurs puissent continuer à se développer et pas aux dépens les uns des autres, il est très important de garder, d'ailleurs, c'est au coeur de l'ADN montagnard, si je puis dire, cet esprit de cordée de solidarité et si je le dis, c'est justement parce que j'ai bien en tête, pour reprendre les statuts de la Caisse des dépôts et consignations, je le cite, que ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'État et les collectivités territoriales après s'agissant du cas que vous évoquez et de la stratégie déployée par la Compagnie des Alpes, il vous a pas échappé que la Compagnie des Alpes, la Caisse des dépôts et consignations, on est actionnaire à hauteur de 39 % c'est donc pas un actionnariat qui est majoritaire et que par ailleurs s'agissant du contrôle de la Caisse des dépôts et consignations, c'est bien le Parlement qui joue aussi un rôle éminent à travers le conseil de surveillance qui, présidé par une parlementaire Sophie errante à qui j'ai pu m'ouvrir d'ailleurs du sujet que vous évoquez sur le nécessaire équilibre à garder et avec 2 membres de la Haute Assemblée, Viviane Artigalas, Jérôme Bascher, donc je pense, vous pouvez saisir également de ce sujet donc je pense qu'il est important, encore une fois et je l'ai dit aux acteurs de la montagne de trouver un bon équilibre et en tous les cas, je serai aux côtés des élus pour continuer à faire passer ce message à l'ensemble des acteurs. Merci. Monsieur Vial, vous avez 18 secondes. merci, monsieur le ministre pour pour votre réponse je ne manquerai pas de solliciter mes collègues mais je pense que le gouvernement a aussi son rôle à jouer, a surtout son rôle à jouer pour vérifier que les les objectifs fixés à cette compagnie correspondent encore aux objectifs politiques d'intérêt général qui avait été fixé, on n'a pas de crainte absolue pour le moment, mais le long, l'enjeu c'est que les profits réalisés sur le théâtre montagne profite au développement de la montagne et notamment aux enjeux de la diversification et et donc qu'on puisse veiller à cela, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à Monsieur Daniel Laurent pour la question orale numéro 1981 au ministre de l'Économie et des finances et de la relance. Madame la présidente, monsieur le ministre, ma question, mes chers collègues, ma question porte sur les conséquences des futures modalités de perception de la taxe d'aménagement pour les ressources des collectivités locales et des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, l'article 155 de la loi de finances pour 2021 à modifier plusieurs articles du code de l'urbanisme relatif à la taxe d'aménagement ainsi les autorisations d'urbanisme délivrées après le 1er janvier 2023 seront exigibles à la date de réalisation définitive des opérations au sens de l'article 1406 du code général des impôts, soit dans les 90 jours à compter de la rivière réalisation définitive des travaux d'aménagement avec ces nouvelles modalités d'État crainte un risque de non-recouvrement de l'impôt en cas d'inachèvement volontaire des travaux ou de non-déclaration d'achèvement des travaux et une diminution des ressources des collectivités locales, de même le passage d'un dispositif de paiement de cette taxe, fondée au 31 décembre 2022 sur la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme un dispositif s'appuyant sur la date d'exigibilité après l'achèvement des travaux au 1er janvier 2023 entraînera pendant une certaine durée, une baisse très importante dans la perception des recettes pour les collectivités, les dans la ressource dépend principalement de la part de la taxe d'aménagement départemental qui leur est dédié, monsieur le ministre, quelles dispositions comptez-vous mettre en oeuvre pour garantir l'effectivité de la perception des recettes dans les conditions prévues selon le nouveau dispositif et quelles mesures d'anticipation, seront prises pour pallier l'impact financier pour les collectivités, les CAUE durant cette période transitoire, je vous remercie pour votre réponse. Merci, la parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du tourisme, des Français de l'étranger de la francophonie et des petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup madame la la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, monsieur le sénateur Laurent alors effectivement un certain nombre d'inquiétudes s'étaient fait jour pendant la la discussion de la loi de finances pour 2021 suite au transfert à la DGFIP de la gestion de détaxe d'urbanisme qui sont aujourd'hui je dirais par les directions départementales des territoires et de la mer, les DDTM, alors je veux dire que pour répondre à la première des inquiétudes, c'est-à-dire le fait que finalement il n'y a jamais de changement faute d'achèvement je veux dire que hé bien les nouvelles modalités de gestion de la taxe ne reposeront pas sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux mais elle deviendra exigible cette taxe au moment de la déclaration à la DGFIP du changement foncier affectant la propriété et c'est une loi qui d'ores et déjà oblige chaque propriétaire a déclaré ces changements dans les 90 jours et donc le nouveau circuit il est fondé sur une obligation fiscale qui est opérationnellement beaucoup plus fiable, effectivement, que les déclarations d'de telle de d'achèvement des travaux, pardonnez-moi, seconde inquiétude c'est celui du décalage de perception des recettes à court terme, ça risque, on a pris très au sérieux, on a voulu le documenter, un rapport à l'Inspection générale des finances et puis également la DGFIP pour estimer l'effet de la réforme sur le rythme de perception des recettes par les collectivités à date au regard de ces éléments, nous considérons que ce risque est faible et toutes les études statistiques confirment l'absence d'impact négatif pour la trésorerie des collectivités locales, parce que tout simplement les délais de traitement sont avec la procédure actuelle substantiellement plus long qu'avec le nouveau circuit, même en tenant compte de l'exigibilité décalé et donc joue pleinement vous rassurer, il y a une ordonnance en cours d'élaboration naturellement à prendre dans les prochaines semaines prochains mois elle va faire l'objet d'une consultation approfondie des collectivités pour apporter toutes les garanties nécessaires visant à sécuriser les ressources fiscales. Si. Monsieur Laurent vous avez 17 secondes. Je n'ai pas besoin de tout ce temps-là, merci Monsieur le Ministre, pour votre réponse, mais surtout ce qui est important, vous m'avez parlé de de l'ordonnance, vous savez qu'il y ait a une campagne présidentielle et un délai qui est fixé pour cette élection, il serait souhaitable que soient prises avant. Merci. La parole est à Madame Hélène Conway Mouret voilà question orale, numéro 2004 au ministre délégué chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie et des petites et moyennes entreprises. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, dans le monde 500 consul honoraire, tous bénévoles, proximité, écoute et sont souvent les premiers interlocuteurs des ressortissants français résidant ou de passage en cas de difficultés financières, maladie, accidents graves, perte et vol, ils sont également un soutien administratif important pour les consulats, notamment pour la remise des titres d'identité établissement des certificats de vie au recueil des procurations de vote, il assure un maillage territorial particulièrement appréciable dans tous les pays et apporte une aide précieuse dans la promotion des Liens économiques et culturels grâce à leur connaissance des acteurs locaux, des relais indispensable pour nos ambassades au vu de l'implication des consuls honoraires je souhaiterais savoir s'il est envisagé de me reconnaître et valoriser leur rôle auprès des ambassades et consulats il pourrait par exemple avoir une adresse courriel standardisée du type prénom Point diplomatie Point gouv Point FR pourraient aussi participer à titre consultatif aux réunions pour l'attribution d'aides d'urgence aux Français vivant dans la région, enfin, afin de faciliter les démarches de nos concitoyens, il semble urgent d'élargir leurs prérogatives en leur donnant la possibilité d'accorder des laissez-passer ou de saisir manuellement des demandes de renouvellement de titre d'identité pour les personnes dans l'incapacité de se déplacer l'heure y compris Monsieur le Ministre, leur engagement et leur dévouement sur le terrain, méritent toute notre reconnaissance et que nous répondions au mieux à leurs demandes. Merci, la parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne Ministre délégué chargé du tourisme, des Français de l'étranger de la francophonie et des petites et moyennes entreprises. Merci beaucoup, madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, sénatrice, madame la ministre Conway Mouret très clairement les consuls honoraires sont là aussi, on parlait de maillon tout à l'heure des maillons très précieux de cette chaîne cet écosystème qui vient en appui à la vie quotidienne de nos compatriotes établis hors de France, 493 agence consulaire en en activité, ce qui permet effectivement un maillage très très étroit et assez unique avec une mission essentielle de protection consulaire d'assistance nos ressortissants connaissons des 10 des difficultés puis aussi naturellement des acteurs précieux de la diplomatie culturelle de la diplomatie économique, bref de l'influence française, on a d'autant plus d'ailleurs dans ces temps de crise pandémique vous le disiez, ils ont un certain nombre de de compétences et vous proposiez qu'ils soient peut-être mieux mises en valeur, je veux dire en terme d'outils que l'idée d'une adresse Mail commune ou identiques, moi je suis tout à fait prêt à la creuser comme nous l'avons fait pour les conseillers des Français de l'étranger, néanmoins, il faut voir que ce sont aussi des personnes qui sont pleinement engagés dans leur vie professionnelle, qui par ailleurs sont connus, souvent au titre de leurs autres engagements et et communique souvent avec leurs propres outils, mais en tous les cas, je, je suis prêt naturellement à à mettre à l'étude cela et et de façon plus globale, parce que, aujourd'hui, effectivement, le décret précise bien ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire le Sénat avait fait en 2005, une étude comparée des statuts des des des consuls honoraires, je trouve que ça aurait de la valeur de continuer à faire un certain nombre de, de, de, de comparaisons internationales et de regarder peut-être ce qui peut nous inspirer, en tous les cas sur le la matière sur laquelle s'est c'est consul honoraire pourrait intervenir avec en tête le fait que ce sont des personnes qui restent bénévoles qui ont aussi beaucoup d'autres activités à conduire et donc il faut veiller aussi à faire en sorte que la charge qui leur interposés soit compatible avec tout cela, pour ne pas décourager naturellement les bonnes volontés, mais vous le voyez donc une ouverture à un travail en tous les cas sur le c'est qu'on sait. Merci, Monsieur le Ministre, merci. Madame Conway Mouret, vous avez 41 secondes. mais écoutez Monsieur le Ministre, c'est la 2ème fois qu'ont répondu de façon très positive à une question orale que que je vous pose la dernière fois c'était en juin 2021, c'était pour la prise en charge totale D. A. S. H dans les lycées à l'étranger, maintenant vous répondez à cette demande, qui est une demande récurrente des consuls honoraires alors c'est vrai qu'il ne faut pas de, de, de, de travail, mais en même temps ils ont des des roquettes et et celle-ci opposé notamment sur le le travail que j'ai pu réaliser avec 3 consul honoraire en Irlande, de Gaulle de Limerick et et de Cork et je pense que l'attribution d'une adresse courriel standardisé nécessaire tant à la reconnaissance du rôle des consuls honoraires au regard des autorités locales que pour des raisons évidentes de sécurité et de protection des données parfois sensibles qu'ils échangent avec les ambassades en tout cas, nous avons tout intérêt à continuer à réfléchir ensemble. merci, la parole est à Madame Laurence Cohen pour la question orale numéro 1947 la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci madame la présidente, madame la ministre, dans le Val-de-Marne, un comité de parents s'est créé, regroupant les villes d'Arcueil, Gentilly, Chevilly-Larue gentil Gentilly l'Haye-les-Roses le Kremlin Bicêtre Rungis et Villejuif et il a recensé 970 enfants et adolescents handicapés sans solution d'accueil et de prise en charge dans des structures spécialisées ou en milieu ordinaire, sur l'ensemble du département, ce chiffre est ce diagnostic constitue concernant sont partagés par la délégation territoriale de l'Agence Régionale de Santé d'une manière générale, l'offre est sous-dimensionné saturé ou inaccessible car hors secteur ces enfants et ces adolescents se retrouvent donc des mois voire des années, en ruptures de parcours sans solution adapter leurs parents contraints de les garder à domicile du coup ben il y a des retards, des régressions dans le développement de ces enfants, faute de professionnels pour les accompagner, malgré plusieurs rendez-vous avec l'ARS du Val-de-Marne, aucune proposition concrète d'accueil n'a pu être mise en place puisque les places n'existe pas alors Madame la Ministre quelles solutions et quels moyens comptez-vous mettre en place en urgence pour la prise en charge de ces enfants et adolescents par l'Éducation nationale et le secteur médico-social afin de mettre fin à ce tournant domiciliaire qui assigne les enfants et leurs parents à résidence merci. Merci, la parole est à madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les sénatrices sénateurs madame la sénatrice oui en effet, les problèmes de solutions pour les enfants handicapés sont au coeur de nos réflexions avec les maisons départementales des personnes handicapées et donc bien sûr avec les présidents de département, avec qui nous partageons cette politique de solidarité et cette politique justement d'accompagnement des parcours, nous avons déployé des équipes mobiles d'appui à la scolarisation justement pour répondre à ces besoins d'accompagnement, ce nouveau dispositif qui favorisent justement la continuité du parcours de l'élève, en apportant un étayage médico-social, aux équipes enseignantes ces équipes mobiles, donc qui sont tenus par les organisations gestionnaires que je salue un dans leur travail justement, de changement de pratiques organisée en réseau départemental sont une ressource précieuse pour soutenir des enseignants et bien souvent, pour permettre aux Antilles en aux enfants handicapés de poursuivre lorsque l'arrêté à l'école à la rentrée 2021 c'est 166 équipes mobiles qui sont déployés, ce sont des nouvelles équipes nous travaillons justement encore à l'accélération pour 2022, en parallèle, nous continuons à renforcer les moyens des associations, cela a donné notamment au déploiement de nouvelles solutions médico-social en 2021, au niveau national, une augmentation de 2600 places de services d'éducation spéciale et de soins à domicile les Sessad nous avons créé 89 class autistes qui ont permis de scolariser 350 enfants supplémentaires dans le Val-de-Marne, puisque vous m'interrogez sur le Val-de-Marne et ce malgré la crise 3 classes autisme des unités d'enseignement maternel autisme ont été créés depuis 2020 de nouvelles classes ouvriront à la rentrée de septembre prochain, l'une pour les enfants autistes, l'autre pour des enfants polyhandicapés et je tiens à souligner cette grande avancée pour que justement la grande différence, les enfants peut dire handicap puce à prendre sur les bancs de l'école avec les autres, ce départ bénéficie également d'une unité localisée d'inclusion scolaire et d'un dispositif d'autorégulation pour les enfants autistes, c'est très transformateurs des pratiques dans l'ensemble de la communauté éducative, par ailleurs, madame la sénatrice afin de prévenir les départs contraints en Belgique, j'ai déployé un plan de 90 millions d'euros pour les régions concernées, pour la première fois, ce gouvernement a préféré agir vraiment, plutôt que de subir ces départs concrètement cela se traduit en Île-de-France par 51 millions d'euros supplémentaires pour construire des solutions nouvelles, au total, il y a 16 projets propres au Val de Marne qui ont été déposés par les associations auprès de l'Agence Régionale

ils sont a suffit, ils ne sont pas suffisamment nombreux en plus, il y a une difficulté de recrutement au niveau des AESH les Ulis ce ne sont pas assez développé et puis ce qui concerne également les places en IME ou au sein des unités d'enseignement maternel autisme, vous l'avez dit, ne sont pas en rapport avec les besoins réels sur le le terrain et ça rend les attentes extrêmement longue, alors je sais que personnellement, vous souhaitez que ces en pour ces enfants garantissent le respect leurs droits et de leur dignité, mais sur le terrain 970 enfants qui n'ont pas, c'est vraiment très grave et c'est un abandon merci nationale malgré les mais le discours sur l'école inclusive.

plusieurs années, se traduisant notamment par des baisses tarifaires de plus en plus drastiques qui mettent en difficulté la continuité de leur l'activité en effet alors que plus de 32000 collaborateurs des PS contribue largement à la mobilisation dans le secteur de santé pour la gestion de cette crise sanitaire anti-participant notamment à libérer des lits d'hôpitaux en organisant de la prise en charge de patients à domicile, plus de 60000 patients Covid ont été pris en charge en oxygène et aux thérapies durant les premières vagues, aucune mesure n'a été prise par le gouvernement pour reconnaître cette profession si les nombreux professionnels de santé ont bénéficié à juste titre d'augmentation tarifaire d'de l'allocation pour l'augmentation de leurs salariés ou encore d'une reconnaissance de leur rôle d'de prestataires de santé n'ont eu aucune et sont les grands oubliés de ces évolutions, le Ségur a été très hospitalo-centrée et le gouvernement doit attend entendre la déception des PSA des et plus globalement de tous les acteurs de santé à domicile en la matière, madame la ministre, quelles mesures compte prendre le gouvernement pour reconnaître les PS AD et leur rôle dans le système de santé merci. Merci, la parole est à madame Sophie Cluzel pour secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci madame la présidente, madame la sénatrice chaque jour les prestataires de services et distributeurs de matériel se déplacent partout en France pour être au plus près des patients, ce service de proximité est essentiel pour notre système de santé, les patients les connaissent et les reconnaisse parce que chacun d'entre nous un moment de sa vie, nous aurons peut-être besoin de de la mobilisation quotidienne ne s'est pas démentie depuis le début de la crise pour apporter aux patients les services dont ils ont besoin, le ministre des solidarités, de la Santé s'est engagé dans ses travaux afin de mener une réflexion sur le rôle de cette profession et sur la méthode pour évaluer reconnaître et tarifée, une prestation, cette étape est indispensable car, aujourd'hui, nous ne disposition, nous ne disposons d'aucun référentiel permettant de décrire et de calibrer les prestations qui sont réalisés le rôle majeur des prestataires et bien d'être aux interfaces entre les différentes professions de santé, en permettant de favoriser le retour à domicile, ainsi que l'autonomie des patients et des personnes en situation de handicap, il s'agit aussi de respecter les responsabilités et les compétences de chacun, je tiens à rappeler que le gouvernement accompagne de longue date, les acteurs de ce système, la dépense moyenne, remboursé de ce secteur augmentent de plus de 5 % par an depuis 2017 en tenant compte aussi des baisses tarifaires cette croissance témoigne du soutien du gouvernement et donc de la valorisation importante de ce secteur pour poursuivre les travaux, nous privilégions le dialogue conventionnel avec les acteurs, en lien avec le comité économique des produits de santé le ministre Olivier Véran lui a d'ailleurs demandé de présenter aux acteurs rapidement ses orientations, problème de 2022 la renégociation de l'accord-cadre doit aussi être un objectif partagé car il est l'acte fondateur d'une nouvelle dynamique pour les prestataires, vous le voyez nous restons attentifs à leur situation. Merci mamie Micouleau 6 secondes merci madame la ministre, pour votre réponse, je pense que les prestataires de santé à domicile apprécieront cette réponse : 1000 demandes, surtout que ce soit conclusif pour eux, c'est-à-dire que, il y a une revalorisation de 2 de leurs mains. merci, cher collègue, la parole est à monsieur Guillaume Chevrollier pour l'action râle N° 2000 59 ans, ministre des solidarités et de la santé. Merci madame la présidente, madame la ministre, 16 métiers du secteur médico-social vont bénéficier d'une revalorisation de 183 euros Net mensuels, quelle que soit leur statut privé ou public, cette initiative est encourageante, mais elle est insuffisante, surtout lorsque on sait que certains ont été oubliés en effet la semaine dernière, j'ai visité la maison d'accueil spécialisée pour adultes handicapés, le Saint Amadou à la seule crâne dans mon département de la Mayenne et les personnels dévoués m'ont interpellé sur l'attribution des revalorisations salariales du Ségur, l'inquiétude est notamment due au périmètre de la réforme car seuls certains salariés du secteur handicap financé par l'assurance maladie, sont concernés par les différentes annonces, cette situation crée d'une part une inquiétude entre les salariés et, d'autre part, un contentieux pour les employeurs des établissements privés solidaire qui, pour le même travail rémunère différemment leur professionnel, le refus de revaloriser de manière identique tous les métiers du secteur médico-social privé non lucratif induit mécaniquement une rupture d'égalité de traitement entre professionnels exerçant un métier dans des secteurs d'activité différents, vous le savez madame la Ministre, le secteur médico-social connaît aujourd'hui en France une crise profonde sans pareil représentant un grave danger pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap, je peux témoigner de l'investissement de ces soignants de ces professionnels éducatifs des psychologues qui font un travail remarquable, ils sont confrontés à des situations douloureuses, ils sont en première ligne, leur travail est essentielle auprès de ceux qui souffrent, donc nous avons besoin de il faut absolument reconnaître leur travail et revaloriser leur salaires alors quelles mesures entendez-vous mettre en place pour rétablir une équité de traitement entre les différents personnels du secteur médico-social à à travail égal, salaire égal pour le même travail pour le même public, c'est une question d'égalité, il est plus que jamais urgent d'agir, et les professionnels compte sur vous. Merci, la parole est à madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, conscient des difficultés rencontrées par les professionnels du secteur social et médico-social, le gouvernement a pris des engagements forts visant à une meilleure reconnaissance de leur engagement dans la continuité de la mission qui a été confiée à Michel Lafourcade, un 1er accord a été signé le 11 février avec l'ensemble des fédérations, employeurs et des organisations syndicales pour revaloriser l'ensemble des personnels non médicaux des établissements sociaux, médico-sociaux rattachés aux établissements publics de santé aux Epad relevant de la fonction publique hospitalière à la demande du gouvernement, Michel Lafourcade ensuite poursuivi des discussions, il a travaillé avec les autres, les organisations syndicales également et les fédérations employeur aujourd'hui. Nous avons décidé de revaloriser les 104 de 183 euros Net les professions que vous avez cité les 16 professions en avance de phase au 1er novembre parce que nous avons entendu justement cette inéquité de traitement pour les mêmes professions nous avons été plus loin 70000 soignants au sens large du terme, les paramédicaux étaient revalorisées en avance de phase au 1er novembre au lieu du 1er janvier 2022, et nous avons voulu aussi faire cette avance dans les établissements relevant des départements pour que, comme vous l'avez très justement dit a même profession il y a cette revalorisation pendant ce temps, les travaux continuent, avec notamment la mission Piveteau, qui travaille sur la reconnaissance de ces métiers de l'accompagnement social et médico-social et comme s'était engagé des fédérations employeur elle continue aussi les travaux de rapprochement des conventions, donc nous ne lâchons rien, nous continuons à travailler, à travailler, nous espérons par la grande conférence sociale qui a été annoncé par le 1er ministre qui se tiendra courant du 1er trimestre de cette, travailler justement à une perspective d'amélioration, avec en même temps, les travaux des fédérations et en même temps, les travaux de la mission Piveteau, donc oui, nous sommes à leurs côtés et nous nous engageons fort pour cette reconnaissance très bientôt. Merci, La parole est à madame Céline Brulin pour la question orale, numéro 2013 au ministre des solidarités et de la santé. Merci madame la présidente, madame la ministre, le service d'urgences du centre hospitalier Caux Vallée de Seine à Lillebonne en Seine-Maritime, a dû fermer à plusieurs reprises ces dernières semaines, faute de médecins son service mobile d'urgence et de réanimation sont SMUR connaît une situation similaire depuis 2019, l'établissement qui ne comptait que quatre, médecin urgentiste a pu en recruter 2 récemment mais il faudrait 12 équivalents temps plein face à ce problème, l'hôpital doit recourir aux intérimaires, qu'on pourrait, pour certains, plutôt qualifiés de mercenaires qui font payer à prix d'or leur vacations grevant d'autant les Budgets de l'établissement, que le gouvernement compte-t-il mettre en oeuvre, face à cette situation, j'ai bien conscience qu'elle n'est pas isolé mais elle se conjuguent chez nous à une pénurie de médecins de ville, ce qui tend à accroître encore évidemment la pression sur les urgences, pourquoi refusez d'encadrer le marché de l'intérim libéral un encadrement qui ne peut pas, d'ailleurs se limiter au seul secteur public car cela renforcerait la concurrence avec le privé, aggravant d'autant la situation actuelle, les 90000 habitants du bassin de vie du centre hospitalier Caux Vallée de Seine et leurs élus craignent légitimement une perte de chance pour les patients, je rappelle, par ailleurs, la présence de nombreux sites Seveso sur notre territoire de même cette une pénurie impact d'autres acteurs du secours, je pense par exemple aux sapeurs-pompiers qui sont de plus en plus appeler sur des interventions qui ne relève pas de leur compétence première et risquent d'être eux-mêmes en difficulté pour leurs autres interventions prioritaires, c'est pourquoi, avec les élus locaux du secteur, nous demandons une affectation prioritaire de médecin au centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine afin qu'il retrouve toute sa capacité d'accueil et de service, je vous remercie. Merci, la parole est à Madame Annick Girardin, ministre de la mer. sur les difficultés démographiques médicale au centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine et en son absence, il m'a demandé de vous lire sa réponse tient une place essentielle sur son sur son territoire au regard bien entendu de la crise sanitaire, la Normandie, comme l'ensemble du territoire national rencontrent des difficultés sur le fonctionnement de certains services d'urgence, vous l'avez dit, afin de pallier ces difficultés, l'ARS en lien avec l'ensemble des établissements publics et et privés disposant d'un service d'urgence et et le SAMU anticipe les tensions pour limiter les suspensions au maximum et y faire face de manière solidaire s'avère dans de très rares cas inévitables alors une équipe territorial d'urgentiste a été mise en place dès 2020, au sein du Groupement hospitalier du territoire dont fait partie le avec un accompagnement financier important, cette organisation était la coopération entre les établissements, en permettant aux praticiens urgentistes exerçant dans l'un des sites du j'ai acheté sur la base du volontariat dans les autres établissements ce dispositif, il sera renforcée, madame la sénatrice par l'application de la prime de solidarité territoriale qui permettra à un praticien temps plein d'exercer, en plus de ses obligations de service sur la base du volontariat, bien sûr, dans un autre établissement de santé que celui auquel il est rattaché, enfin, l'article 33 de la loi dite Rist visant à améliorer le système de santé prévoit, comme vous le savez, un contrôle renforcé de l'intérim médical après échange avec les acteurs du système de santé concernés, les représentants professionnels et les syndicats le Ministre de la Santé a décidé que la mise en oeuvre et de la réforme se ferait en 2 temps si la cartographie précise de la situation actuelle de l'intérim médical sur le territoire a été réalisée l'application stricte de la réforme se fera plus tard dans l'année, par ailleurs, la réforme de l'accès à une étude aux études médicales, avec la suppression du numerus clausus permet d'augmenter le nombre de professionnels en formation assis à Caen et à Rouen, il y a environ 20 % d'étudiants dans des études médicales de plus qu'en septembre 2021 les places que vous évoquiez, Madame la Ministre, ce sont les étudiants en médecine qui se sont battus et qu'on s'qui ont saisi le Conseil d'État pour qu'elle soit ouverte parce que votre collègue, Madame Vidal s'y refusait, je crois qu'il est en effet urgent de former des médecins, parce qu'en Normandie parmi les spécialités qui manque énormément, il y a précisément les urgentistes et je crois qu'il faut développer un grand effort de formation dans notre région en particulier, merci, merci, cher collègue. Alors. La parole est à monsieur le questeur Jean-Pierre Sueur pour la question orale numéro 1998 au garde des Sceaux, ministre de la justice. Merci madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je voulais appeler votre attention et j'ai appelé l'attention bien sûr du garde des Sceaux, comme vous le savez, sur l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 2021 cet arrêt concerne le 1er cas de mise en examen en France, dans le cas de la compétence universelle en matière de films de guerre et de crimes contre l'humanité. La Cour de cassation a considéré que l'accusé ne pouvait être poursuivi en France pour crimes contre l'humanité car cette notion n'existe pas dans le droit pénal syrien. Je voulais vous appeler Madame la Ministre, que le Sénat a adopté une proposition de loi portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale qui avait pour effet d'élargir va compétences territoriales des magistrats français afin qu'il puisse poursuivre et juger les auteurs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à l'étranger, le gouvernement a finalement donné un avis favorable en 2019 lors du débat sur le projet de loi relatif de programmation et de réforme de la justice, un amendement ayant pour effet de supprimer ce verrou de la double incrimination mais en le limitant au génocide, cet amendement a été adopté, inscrit dans la loi, malheureusement. permis, tout n'a pas pris en compte les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité alors ma question est très simple, vous voyez que cette double incrimination supposerait que notre droit fut identique à celui de pays qui ne relèvent pas des mêmes valeurs démocratiques qui sont les nôtres, merci, cher collègue, et donc je voulais vous demander, non, non, merci, Charles, oui, oui, mais vous savez bien compris Madame la Ministre, si vous allez lever ce verrou, je vous remercie. Merci beaucoup, la parole est à Madame Annick Girardin, ministre de la mer. Le présidente mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le le le sénateur Jean-Pierre Sueur veuillez excuser mon collègue Éric Dupond-Moretti pour son absence, il m'a demandé donc de vous lire sa réponse la France dispose depuis la loi du 9 août 2010 d'une compétence juridictionnelle en matière de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, instaurée par l'article 689 11 du code de procédure pénale, les juridictions françaises peuvent ainsi déclencher des poursuites à l'encontre une personne soupçonnée de ces crimes, dès lors qu'elle réside habituellement en France sous la réserve qu'aucune juridiction internationale ou nationale ne demandent la remise ou l'extradition de la personne, dès lors que ces faits et, à l'exception du génocide depuis la loi du 23 mars 2019 sont également puni dans l'État étranger où ils ont été commis, sauf si le dit État est parti de la Convention sur la Cour pénale internationale dès son arrêté, le 24 novembre 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a interprété l'exigence de cette double concerne une heure la procédure ayant donné lieu à cet arrêté concerne un ressortissant syrien, vous l'avez dit, entrée sur le territoire français en 2015 mais en examen du chef de complicité de crimes contre l'humanité, la Cour de cassation a jugé, s'agissant des crimes contre l'humanité que l'exigence posée par le code de procédure pénale, selon laquelle des faits et doivent être punis par la législation de l'état où il a été commis inclut nécessairement l'existence dans cette législation d'une infraction comportant un élément constitutif relatif à une attaque lancée contre une population civile en exécution d'un plan concernés,

qui constituent effectivement et qui sont à l'origine de cette poursuite dans l'affaire qui a été, qui a été saisie, alors il n'appartient pas et Emmanuel Ferry astre, monsieur le sénateur au gouvernement de faire des commentaires, les conséquences de cette décision sur les procédures ouvertes des chefs de crimes contre l'humanité, crimes de guerre sont en cours d'évaluation. je vais vous dire une chose, tout le monde, c'est le temps qu'il a, que ce soit vous les sénateurs et les ministres en plus monsieur que ça, vous êtes arrivé vraiment la limite ici, on a plusieurs collègues là qui arrive en retard et nous, ici, à la séance, on est obligé de gérer, sincèrement, j'ai jamais vu une chose comme ça. C'est un rappel au règlement, madame la présidente, je fais un rappel au règlement

pour venir, elle, je pensais que je passer dans un quart d'heure, donc je ne me suis pas occupé du tort ni de rien, je me suis occupé de la question de savoir que s'il faut que notre droit, soit le même que le droit syrien pour punir les crimes contre l'humanité, c'est quelque chose d'inacceptable, je leur ai dit et je vous remercie de me l'avoir de m'avoir permis de le dire, madame la présidente. Bien, bien sûr, je ne nie pas là l'intérêt de de votre question, bien entendu, mais moi j'ai à gérer aussi aussi le temps mais acté donné bien sûr de votre rappel au règlement, merci, la parole est à Madame, Mélanie Vogel pour la question orale numéro 1973 transmise à la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes de la diversité et de l'égalité des chances. Merci. Si cher collègue, Madame la Ministre, l'adoption de la de la loi relative à la bioéthique du 2 août dernier fut, vous le savez, une victoire historique dans la lutte pour l'égalité entre toutes les femmes, l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules signifia ce jour-là que pour d'innombrables française, la perspective de fonder une famille ne devait plus être synonyme de procédures interminables, j'ai donc suivi attentivement la mise en oeuvre de cette loi, notamment pour nos concitoyens établis à l'étranger que j'ai l'honneur de représenter et je dois dire que je suis assez frappé par sa lenteur, au moment où j'ai déposé cette question, c'était en décembre les instructions de la circulaire de présentation des dispositions relatives à la loi du 2 août n'était toujours pas transmise au consulat, il aura fallu attendent plus de 3 mois entre la publication de la circulaire et les instructions transmises au consulat, ce sont maintenant 6 mois depuis l'adoption de la loi pendant ces 6 mois,

moi, me direz-vous peut-être que c'est un délai raisonnable pour qu'une nouvelle loi soit appliquée, mais aujourd'hui les familles concernées sont obligés de passer par une transcription de l'acte de naissance du pays où elles habitent transcription qui dure en moyenne 3 mois pour les couples hétérosexuels, mais qui peut durer jusqu'à 18 mois pour les couples homosexuels pour toutes les familles qui n'ont pas pu établir d'acte de naissance français avec la double filiation depuis deux août ça peut donc être 2 ans d'attente, au total, il n'est pas clair non plus, si le nom de famille figurant sur l'acte de naissance étrangers sera opposable pour l'état civil français ou si les familles pourront choisir pour leur enfant le nom de leur choix, comme le prévoit le code civil, il serait incompréhensible que ces familles soient pénalisés, donc ma question est la suivante : quelles mesures sont prévues pour que ces familles puissent obtenir le plus rapidement possible inscription de leur enfant à l'état civil français avec le nom de leur choix, un prolongement du délai légal de 30 jours est-il envisageable, et sinon, est ce que ce processus. L'état Madame Annick Girardin, ministre de la mer. Madame la la sénatrice Mélanie Vogel, je vais vous lire la réponse de mon collègue Éric Dupont-Moretti, je me réjouis comme vous des dispositions que de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique qui a notamment ouvert l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées, l'article 342 11 du code civil issu de cette loi dispose que pour les couples de femmes ayant recours à une assistance médicale à la procréation postérieurement à la loi, reconnaissance conjointe peut-être faites devant le notaire en même temps qu'est donné le consentement à l'assistance médicale de procréation avant que le processus procréatif il faut distinguer la situation des actes de naissance étrangers transcrit et celle des actes de naissance, dressé par les postes consulaires lorsqu'il a été dressée à l'étranger par une autorité étrangère, l'acte de naissance de l'enfant issu d'une assistance médicale à la procréation, réalisé par un couple de femmes peut-être transcrit totalement sur les registres de l'état civil français si la étrangers et régulier exempt de fraudes et établi conformément au droit de l'État étranger le couple de femmes n'a pas à produire de reconnaissance conjointe anticiper ou de reconnaissance conjointe pour obtenir la transcription totale de l'acte de naissance étrangers sur le registre de l'état civil français, ces différences, ces différents pardon lorsque le poste consulaire français établi, l'acte de naissance de l'enfant né à l'étranger, les nouvelles dispositions introduites, vous l'avez dit, par la loi, sont applicables et le couple de femmes devra produire une reconnaissance conjointe anticiper les postes consulaires ont été informés de ces nouvelles dispositions, il ne devrait pas avoir de difficultés à enregistrer les naissances dans le délai de 30 jours prévu par la déclaration des enfants nés à l'étranger en particulier hors Europe, enfin, la loi relative à la bioéthique a introduit des dispositions particulières sur le choix du nom de famille de l'enfant, le couple de femmes qui a eu recours à une assistance médicale de programmes à la procréation et qui a établi une reconnaissance conjointe anticipée peut choisir le nom de famille dévolu à l'enfant soit le nom de l'une d'elles, soit leur donnant accolés dans l'ordre choisi par elle, dans la limite des noms de famille pour chacune d'elles, cette facilité est également ouverte mais ça va à l'étranger. la parole est à Madame Frédérique Espagnac pour la question orale, numéro 2 1038 à la ministre de la mer. des quotas de pêche et pour les poissons plats que la baisse est la plus conséquence une baisse de 36 % des 2022, c'est une catastrophe pour de nombreux professionnels basque landais et Girondins, pour la plupart des pêcheurs du Golfe de Gascogne, la seule, c'est 50 % de leur chiffre d'affaires, si on enlève 36 % de ces 50 cela fait quand même un sacré trou d'autant plus que pour les patrons de presse, les pertes iront au-delà du poisson plat quand il pêche un kilo de Sol il pêche aussi un kilo de poisson d'hiver, dont certains ne sont pas soumis à des quotas, donc ils vont perdre également 36 % de ces poissons d'hiver, c'est le coup de grâce pour beaucoup d'entre eux, les directeurs de port du pêche du littoral se disent eux aussi très inquiets sol représentent pour certains, la moitié du chiffre d'affaires de la criée, ils estiment les pertes entre 1,5 et 2 millions d'euros s'il y avait eu une baisse s'il savait qu'il y aurait une baisse, il pensait qu'elle serait l'issue sur plusieurs années la ils n'ont pas d'issue de secours, même si des aides compensatoires devrait être versée sur le fonds européen sur le fait, en plus, les directeurs du crier n'ont aucune assurance et ne savent pas, à ce jour six seront inclus dedans, concernant les pêcheurs si le montant n'est pas à la hauteur de nombreuses exploitations seront en danger en effet selon un pêcheur l'usure, le montant de ces aides promises par l'Union européenne n'est pas fut suffisant pour compenser les pertes, certes ils sont rassurés aujourd'hui on leur propose 70 % de leur chiffre d'affaires journalier néanmoins le calcul des aides par sur une mauvaise estimation des frais fixes, il manque 15 % pour que ces aides soient tant fait acceptable, madame la ministre, je souhaiterais donc savoir je vous demander quels seront les montants des indemnisations versées au titre du film pour les pêcheurs et les criées si les coûts fixes seront pris en compte à leur juste valeur, et si le décret portant sur ces compensations incluant délai de paiement de ces aides, enfin, si le gouvernement va diligenter une étude afin de comprendre les causes de cette évolution du nombre de sol dans le dans la zone du Golfe de Gascogne afin d'oeuvrer en faveur du plus d'une plus grande durabilité de cette espèce. Merci, merci n'à parole est à Madame Annick Girardin, ministre de la mer. Madame la sénatrice Frédérique Espagnac, vous avez raison, à Bruxelles, le 13 décembre dernier 3 sujets importants pour le Golfe de Gascogne : d'abord le bar ensuite effectivement le lieu jaune et la seule d'abord le quota de bar espèce à forte valeur ajoutée pour laquelle j'ai obtenu une augmentation doit être repréciser ensuite pour le lieu jaune, une baisse de 20 % devait être prévu, nous sommes sortis avec une reconduction du quota il y a aussi des points positifs à cette rencontre de décembre à Bruxelles, la seule malheureusement avec un résultat décevant n'est prévisible, puisque le plan de gestion signée en 2019, avec l'accord de de la filière est connue de tous, d'ailleurs, prévoyait une baisse automatique Automatic de 37 %, compte tenu de l'état du stock à partir de là, il a dû, et j'ai dû négocier effectivement l'accompagnement de la pêche je sais combien les efforts demandés aux pêcheurs sont importants, mais je ne peux pas vous laisser dire que rien n'a été fait, vous savez, avec eux, avec eux, en juillet dernier, nous étions réunis à à à Royan, nous avions lancé un groupe de travail décider des arguments que nous allions utiliser à Bruxelles, d'une part, pour essayer de faire que l'automaticité soit pas mises en vigueur, mais ça a pas été possible et d'autre part parce que c'est comme ça, c'est une règle, mais ça a été posée, c'est pas moi qui l'ai signé et les professionnels, on était et était partant, et d'autre part surtout d'avoir un plan d'accompagnement, et c'est là le plus important, bien entendu, ce plan d'accompagnement, financé par le pas ce plan est traduit, il se traduit par la mise en place d'un dispositif d'arrêt temporaire co-construit avec les professionnels, on a souhaité que les conditions soient très large les plus généreuses possible et vous pourrez le constater avec les pêcheurs, soit quand ils sont effectivement très touché, même d'ailleurs jusqu'à 10 de leur valeur totale qui serait effectivement touchées, on a souhaité également que ce soit réactif et que ça puisse couvrir la totalité de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, vous avez parlé de la filière avale, elle est toujours une préoccupation également pour moi, elle pourra être épaulés par des mesures de plus long terme cette fois des mesures d'investissements du plan de relance et du faire la question de l'état écologique, la réponse sera apportée dans le travail que nous menons sur le plan durable pas. Merci madame monstre. La parole est à monsieur Stéphane ce pour la question orale numéro 1590 à la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Merci, merci, madame la présidente, madame la ministre, la mise en oeuvre et de la réforme des études de santé issu de la loi de juillet 2019 devait conduire, d'une part à diminuer le taux d'échec des étudiants en supprimant le numerus clausus dans l'objectif de former 20 % de médecins supplémentaires et, d'autre part à diversifier leur profil et faciliter la réorientation en cas d'échec, l'année 2021 a laissé, a laissé apparaître une réalité bien différente avec des situations dramatiques pour nombre de jeunes de familles nous conduisant au final à augmenter le nombre de places en 2ème année pour tenir compte des redoublements en anticiper chaque université aurait dû augmenter ses capacités d'accueil de 30 % en fait il n'en a rien été, cela a d'ailleurs conduit le Conseil d'État a annulé 2 articles de votre arrêté à l'été 2021 15 universités sur 31 n'ayant pas respecté les augmentations d'accueil des étudiants issus du là c'est du passe, dont celle de Clermont-Ferrand, les victimes sont nombreuses jeunes laissés pour compte, famille, passant de la fierté à l'angoisse inéquité, d'accroissement des numerus clausus selon les universités territoires devenus de vrais déserts médicaux et qui sont condamnés à le rester patient cotisants spoliés, je pourrais élargir ma question aux IFSI mise à mal, elle aussi, par Parcoursup alors que nous avons plus besoin que jamais, d'infirmiers, Madame la Ministre, comment, faute d'avoir anticipé allez-vous infléchir ses injustices pour nos étudiants, je vous remercie. Merci, la parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Merci madame la présidente mesdames et sénatrices, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Sauterel, vous l'avez rappelé cette réforme, elle avait pour objectif de supprimer le numerus clausus et de transformer profondément c'est ce qui a été fait, monsieur le sénateur avec 2663 places supplémentaires créés dans l'accès aux études de santé et 1812 places supplémentaires spécifiquement créée dans le cadre de l'accès aux études de médecine, vous parlez de redoublement, c'était bien une partie du scandale puisque les étudiants réussissent leur année raté leur concours a été obligé de redoubler, ce qui a changé avec cette loi, c'est que les étudiants qui réussissent leur année continue dans leur cursus et on leur 2ème chance à la fin de leur 2ème, année de l'essence : vous parlez des déserts médicaux et de la difficulté à former nos jeunes dans l'ensemble des territoires, c'est exactement la raison pour laquelle, Monsieur le Sénateur, nous avons créé 40 457 licence accès santé répartis partout sur le territoire, y compris dans les universités qui ne comportait pas d'UFR Santé de manière à ce que l'on puisse démarrer ses études de médecine, partout sur le territoire et la réforme du 2ème et du 3ème cycle vont nous permettre d'accueillir là encore plus d'externes plus d'internes partout sur les territoires grâce à sa mise en place, alors oui, tout n'a pas été simple, vous l'avez rappelé la mise en oeuvre a été compliquée par la crise sanitaire, mais nous avons mis en place des ajustements avec une mission d'inspection générale qui a fait des recommandations, un arrêté était est en préparation pour donner suite justement à ce rapport de l'Inspection générale, un comité de suivi local a été installé dans chaque université et un calendrier de rencontres a été établi pour poursuivre à la mise en place de la réforme avec les étudiants, Kant, au nombre de places dans les IFSI, monsieur le sénateur, je ne peux que partager votre opinion, mais les IFSI dépendent des régions, j'imagine que vous ne l'ignorez pas. Merci, la parole est à monsieur arrête pour 33 secondes. Merci, Madame la Ministre, pour ces ces réponses, je je n'ignore pas non plus le contexte de la crise sanitaire, mon mari, ma question avait été posée au mois de mars dernier, donc elle est un peu sur les ici, ce n'est pas la gestion des établissements que je mettais en cause c'était l'orientation via Parcoursup vers les IFSI qui aujourd'hui prive de de ces établissements de certains étudiants, enfin je je veux quand même souligner qu'aujourd'hui des disparités existent de manière très forte dans le numerus clausus selon les universités et que le nombre de médecins généralistes formés pour 100000 habitants en région Auvergne ou dans l'Hérault, dans les Alpes-Maritimes, demeurent très différents et ce qui explique les conséquences. Sur nos territoires, merci, la parole est à monsieur Jean-Pierre Moga pour la question orale numéro 1921 la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Merci madame la présidente, madame la ministre ma question concerne les règles prudentielles de trésorerie des opérateurs de recherche qu'il s'agisse de la loi du 24 décembre 2000 owen de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, des crédits de la mission enseignement supérieur et recherche du budget de l'État ou des crédits du plan de relance prévu de constater que s'ils n'ont pas produit de choc budgétaire en faveur de la recherche, néanmoins ils étaient à j'était attendue et sont les bienvenus. Par ailleurs. Depuis 2 ans avec la commission des affaires économiques du Sénat, j'attire l'attention sur les règles prudentielles excessives provenant de la comptabilité publique et pesant sur la trésorerie des opérateurs de recherche. De telles règles prix veut en effet la recherche française de centaines de millions d'euros de financements qui serait pourtant eux aussi les bienvenus, c'est en particulier le cas d'une norme obligeant a provisionné une somme correspondant à la totalité des comptes épargne-temps et quand j'ai payé comme s'il était demandé, en même temps par tous les collaborateurs. Cette norme n'est pas adapté aux organismes de recherche. Pour des sommes de bénéficiant aucunement à la recherche, il conviendrait donc de l'ajuster pour financer les dépenses de prix maturation des recherches interdisciplinaires et davantage de postes de doctorat ainsi, je souhaiterais qu'une information précise soient communiquées par le gouvernement aux parlementaires sur le niveau de trésorerie détenue par les grands opérateurs de recherche afin d'évaluer le manque à gagner de la recherche française. Pouvez-vous, Madame la ministre me donner des informations relatives à des assouplissements des normes prudentielles en question, comme vous y étiez engagé lors d'une audition devant la commission de la culture en 2020. Merci, la parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Merci madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Jean-Pierre Moga, je partage votre analyse sur le fait que les règles prudentielles sont effectivement parfois très contraignantes et d'ailleurs, un décret financier est actuellement en cours de préparation pour accompagner la modernisation de la gestion des opérateurs de de mon ministère la question de la comptabilité des normes de prévisions sur les différents dispositifs RH que vous mentionnez pourra être envisagée dans ce cadre, les travaux d'instruction à ce sujet sont déjà en cours, comme vous le savez, la masse salariale des oeufs PST comptabilisés or titre de à l'instar de l'ensemble des opérateurs de l'État et cela nécessite donc un cadre rigoureux pour leur donner tous les leviers pour piloter leurs dépenses RH, s'agissant de la trésorerie des organismes de recherche et des oeufs PST si vous souhaitez évidemment mon ministère vous transmettra l'ensemble des données en tant que rapporteur pour avis des crédits de la mairesse pour la commission des affaires économiques du Sénat, vous auriez naturellement plus les demander, dans le cas du traditionnel questionnaire budgétaire annuel adressé par le Sénat à mon ministère, c'est ce que je ce à quoi je m'attendais, mais comme le débat budgétaire n'a malheureusement pas pu avoir lieu en séance publique, devant la Haute Assemblée, hé bien, nous n'avons pas été saisi de cette demande, vous avez raison de de rappeler ce qu'a apporté la loi de programmation pour la recherche, c'est un un véritable choc budgétaire et c'est pour la première fois une garantie de financement après des années de gel de l'effort de l'État en matière de recherche plus d'une dizaine d'années 19 milliards d'euros devaient être engagés suite à la loi Goulard de 2006, mais ça n'a pas été porté par le gouvernement Fillon de de vous renvoyer à ce qui n'a pas été fait il y a 10 ans, je vous remercie et je remercie la la haute assemblée, d'avoir permis en votant cette loi de réarmer notre ruche. Merci, la parole la parole est à monsieur Ronan Le Gleut pour la question orale, numéro 2 1048 transmise à la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Merci madame la présidente, madame la ministre, dans 2 jours, le 20 janvier Les lycéens vont s'inscrire sur Parcoursup qu'ils soient lycéens sur le territoire national ou bien lycéens français à l'étranger. Or, les statistiques du ministère de l'enseignement supérieur qui ont été notamment publié dans un article du journal Le Monde 2 septembre 2021 montent que les les lycéens français de l'étranger sont souvent évincé par Parcoursup, ces statistiques sont révélatrices : le 27 mai 2021 seuls 20 % des 25000 lycéens français à l'étranger, avait reçu une proposition d'admission, contre 54 % des autres lycéens, le 16 juillet 2021, au moment de la la fin de la phase principale d'admission 48 % de ces lycéens français à l'étranger avec une réponse positifs contre 89 % pour les lycéens français français sur le territoire national ou dans le réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, or tous les toutes les familles françaises à l'étranger ne peuvent pas scolariser leurs enfants dans l'un des 545 lycées français à l'étranger, et ce pour 2 raisons principales, la 1ère c'est que quand on habite à des centaines de kilomètres du prochain lycée français, voire même plus demi-kilomètre, je pense au Brésil à la Russie à l'Argentine à l'Australie, hé bien ce n'est pas possible 2ème raison, c'est le coup quant à la scolarité coûte plusieurs milliers d'euros évidemment ce n'est pas possible, donc nous avons cette difficulté et donc les enfants passent leur Baccalauréat dans le système national ou dans un système du type binational Abibac Bachy bac ils abattent par exemple avec l'Italie et donc ma question est la suivante : des collègues parlementaires vous ont interrogé sur ce sujet dans des questions écrites aussi bien députés ou sénateurs au mois de septembre et d'octobre dernier et donc dans 2 jours, l'inscription va avoir lieu pour Parcoursup avez-vous régler cette question afin que les Français de l'étranger soit vraiment considérés comme des Français à part entière et non pas comme des Français à part merci madame la ministre. Merci, la parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, avant que vous prenez la parole et je crois qu'il y a un souci avec le le déroulé que vous voyez mais ne vous inquiétez pas, vous êtes bien sur la liste, excusez-moi, madame la ministre, c'est à vous. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, le nos ministères, celui en charge de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement supérieur accorde évidemment une très grande attention à tous les candidats français dans le cadre de la procédure d'accès à l'enseignement à l'enseignement supérieur Parcoursup quelle que soit leur lieu d'études ou l'établissement fréquenté, c'est environ 25000 lycéens et étudiants scolarisés en qualité de lycéens ou d'étudiants à l'étranger en dehors d'un établissement du réseau de la EFE qui candidate chaque année sur Parcoursup et sur ce total de 2 candidats, ceux qui n'ont pas suivi de scolarité française et non pas le Baccalauréat français sont un peu moins de 4000 chaque année, le taux de propositions reçues par ces candidats et de 82 % in fine et ce qui est tout à fait comparable à la moyenne nationale, compte tenu de la diversité des baccalauréats étrangers considérés, mais vous avez raison dans le temps, les choses se déroulent de façon différente, nous avons donc permis la prise en compte de la spécificité de la formation des élèves ayant suivi sa scolarité étrangère avec la possibilité pour les formations de télé verser les bulletins scolaires correspondant à la scolarité étrangères d'autoriser les bulletins d'un autre format que la notation sur 20 le candidat peut sélectionner le format au moment où il renseigne, c'est notre note sur 5 sur 10 sur 100 notation abaisser le parcours des candidats bilingues et évidemment bien souvent considéré considéré comme un atout pour l'entrée dans les études supérieures, la procédure de préinscription et et la comité d'accès à l'enseignement supérieur est évidemment ouverte à ces candidats, mais c'est vrai que ça prend un peu plus de temps parce qu'ils doivent expliquer le système de formation dans lequel ils sont inscrits, mais cet accompagnement prodigué par ces commissions d'accès à l'enseignement supérieur se fait évidemment au bénéfice de l'ensemble de nos concitoyens, je vois bien. Merci, la parole est à monsieur Laurent Somon pour la question orale numéro 1925 au ministre de l'Éducation nationale de la jeunesse et des Sports. Madame la ministre, que l'État veuille optimiser la gestion des personnels d'accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH et permettre à un maximum d'enfants, d'avoir un accompagnement, cela est très louable à la condition d'répondent aux besoins des élèves en situation de handicap et de proposer au personnel à AESH comme à ED, la reconnaissance qu'il mérite sinon l'État mène une politique d'habillage qui ne satisfait en rien, et comme en cette rentrée 2021 35000 élèves vulnérables n'ont pas bénéficié d'AESH et même à cette rentrée en janvier encore 40 d'entre eux, dans la Somme, n'en bénéficient pas, le recrutement de 4000 nouveaux AESH et l'augmentation des salaires de 600 euros brut par an, issus du budget 2022 ne sont toujours pas à la hauteur des besoins en termes de conditions de travail avec l'ubérisation du métier infligée par les pial notamment en milieu rural avec les déplacements qu'ils imposent des rémunérations sous le seuil de pauvreté, avec une moyenne de 760 euros, une précarité de l'emploi avec des CDD renouvelable pour un an la USH est chargé de l'accompagnement de la socialisation de la sécurité de l'aide à la scolarisation en six tue des enfants en situation de handicap dans la classe pendant le temps scolaire et tout le temps de l'école cette charge requièrent une compétence élargie, donc des formations, les AESH vers l'humain et le bien vivre ensemble, madame la ministre, qu'en est-il de la création d'un véritable statut de la fonction publique pour les AESH et les de la reconnaissance de l'institution dont ils dépendent, dans la Somme, comme partout en France, il n'y a pas de réussite sans accompagnement, d'autant plus que lorsque la compagnie est en situation de handicap, l'éducation nationale doit donc suivre la notification de MDPH, quelle est la réalité de l'inclusion scolaire en 2022, est ce que la MDPH peut administrer son budget et les notifications sont-elles à cette date, toutes satisfaites. Merci, la parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Merci madame la présidente mesdames et sénatrices, messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, saumon, je vous prie d'excuser l'absence de mon collègue, qui m'a transmis cette réponse, vous le savez, l'école de la République est une école qui doit être attentive à chacun de ses élèves et capable de les accueillir tous et c'est pourquoi la scolarisation des élèves en situation de handicap a été une priorité de ce gouvernement qui a souhaité créer un véritable service public de l'école inclusive ces 400000 élèves en situation de handicap accueillis à l'école, c'est presque 20 % de plus en 5 ans, c'est 120000 AESH recruté avec un statut plus protecteur et j'y reviendrai, c'est 1000 300 Ulysse, créer 250 structures spécifiquement dédié à l'autisme, sur l'ensemble du territoire, c'est des familles mieux écoutés, mieux accompagner avec un numéro unique d'écoute des services départementaux dédié les entretiens pédagogique en amont de la rentrée, c'est une organisation territoriale qui a été entièrement repensé, qui s'appuie sur les pôles inclusifs d'accompagnement personnalisé pour paramètre, la coordination des moyens au plus près des territoires et une coopération renforcée avec le secteur médico-social, parallèlement au au recrutement de ces nouveaux avez que j'ai évoquais nous avons pour répondre à la demande et MDPH conduit une action sans précédent de sécurisation des parcours, les contrats aidés ont été transformés en CDD, qui eux-mêmes peuvent déboucher sur des CDI, la rénovation du cadre de gestion qui a permis d'augmenter la période de travail de référence et depuis septembre 2021 une grille indiciaire revalorisé, avec une progression automatique tous les 3 ans, c'est 56 millions d'euros qui sont ainsi mobilisés et enfin le premier octobre, une nouvelle étape qui a été franchi avec un début de gris porté à un indice 341 au-dessus donc du niveau du SMIC c'est une augmentation de 9 points d'indice en début de carrière, alors je vous savez bien sûr sensible à la défense de nos services publics, celui de l'école inclusive, c'est plus de 3,5 milliards de madame la Ministre, 66 % de hausse depuis 2000. Monsieur, vous avez 16 secondes. Rapidement pour dire Madame la ministre effectivement que l'attractivité de ces métiers et la clé de la réussite, je dirais, de cette inclusion des enfants handicapés dans nos écoles, il faut y travailler à la fois sur la formation et la et leur rémunération augmenter de ces personnels. Merci, la parole est à Madame Elsa Schalke pour la question orale numéro 1980 au ministre de l'Éducation nationale de la jeunesse et des Sports. Merci madame la présidente, madame la ministre ma question porte sur les modalités de financement des accompagnants des enfants en situation de handicap au sein des structures périscolaires, nous avons tous à coeur de mener une politique inclusive inclusive pour les enfants en situation de handicap et d'être aux côtés de ses enfants et de leurs familles, pour ce faire, nous le savons, la question de l'accompagnement et centrale, nous vous interpellons régulièrement au sein de cet hémicycle sur le manque d'accompagnants d'élèves en situation d'handicap qui demeure encore actuellement bien trop fréquents, encore récemment j'ai été interpellé par la mère d'articles sème dans le Bas-Rhin, sur ce sujet actuellement dans le sud du département, ce n'est pas moins de 80 élèves qui sont toujours dépourvues, à ce jour d'AESH ce matin, je souhaite également relayé la motion d'urgence prises par la communauté de communes du canton d'Erstein dans le Bas-Rhin, en décembre dernier sur la question du financement dans les temps périscolaires, il apparaît que, suite à une décision du Conseil d'État du 20 novembre 2020, le financement des AESH pendant le temps périscolaire et notamment pendant la pause de midi, doit désormais être pris en charge par les collectivités territoriales et non plus par l'État, suite à un courrier de l'Académie, au mois de septembre des maires du Bas-Rhin et des présidents de communautés de communes mon alerter sur les difficultés engendrées par une telle décision pour une application immédiate au 1er janvier de cette année, il s'agit d'une charge financière et logistique très conséquente pour les collectivités qui sont déjà éprouvée fortement budgétairement, du jour au lendemain des collectivités ont dû repenser toute l'organisation de l'accompagnement de ces élèves, entre le temps scolaire et le temps périscolaire dans des délais très courts, juste avant les vacances de décembre afin que tous puissent se passer au mieux, elles ont dû s'organiser avec les AESH ayant accepté de poursuivre leur mission, madame la ministre, face à l'inquiétude des élus locaux, pouvez-vous nous indiquer si les collectivités devront effectivement prendre en charge et recruter les AESH et si oui, comment votre gouvernement, explique-t-il, un tels changements sur une question centrale : je vous remercie. Merci, la parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Merci madame la présidente, madame la sénatrice, messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, elles achètent la scolarisation des élèves en situation de handicap est une priorité que nous partageons et et c'est un enjeu qui doit évidemment nous rassembler, vous mentionnez la décision du Conseil d'État de novembre 2020, je tiens à apporter quelques précisions cette décision allait clarifier la question des modalités de prise en charge financière de l'accompagnement humain des élèves en situation de handicap dans le cadre des activités périscolaires notamment de restauration par les collectivités territoriales et le Conseil d'État a jugé qu'il appartenait aux collectivités territoriales, et non pas à l'État de prendre en charge l'accompagnement des enfants en situation de handicap lorsqu'elles organisent un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires et périscolaire, cette décision a clarifié le droit existant n'a pas à proprement parler modifié ce droit, mais depuis cette décision évidemment les les services du ministère de l'Éducation nationale travaille à sa mise en oeuvre avec un seul objectif : garantir la continuité de l'accompagnement de ces enfants et pour que cette décision s'applique, il ne faut pas entraîner de rupture pour ces élèves, c'est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale travaille notamment avec le ministère de la cohésion des territoires autour de différents dispositifs mis a mis à disposition, entre l'employeur, le ministère est une collectivité emplois Directs des AESH possible par une collectivité dans le cadre d'un cumul d'activités recrutement conjoint par l'État et une collectivité territoriale et cette décision représente une double opportunité, celle pour les élèves d'avoir un accompagnement de qualité continue sur l'ensemble des temps de la journée et celle pour les AESH qui le souhaitent de compléter leur temps de travail puisqu'on on l'évoquait la grande majorité sont en en travail partiel, les services du ministère se tienne à disposition des collectivités pour travailler toutes ces possibilités, avec comme seule ambition toujours mieux accompagner les élèves en situation de handicap et leurs familles, je suis en mer. Merci madame la ministre, la parole est à monsieur Jean-Marie Mizzon pour la question orale numéro 1915 au Ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, bonjour, je souhaite vous interroger sur la méthanisation à l'origine de ce ce procédé innovant devait permettre des fermes de valoriser leurs propres déchets voir ceux des fermes voisines il présenter des qualités, économique, écologique et énergétique indiscutable aujourd'hui dans certains départements, en Moselle, notamment on constate dans ce domaine, une évolution qui pose question, en effet, certains agriculteurs ne cultivent plus pour nourrir les hommes ou les animaux mais pour alimenter le seul méthaniseur plantant des dizaines voire des centaines d'hectares de serres de céréales : du maïs notamment dans ce seul but, si ce mouvement devait se poursuivre, il pourrait être même sans aller jusqu'à sa généralisation avoir pour conséquence de télescoper à terme notre volonté de souveraineté alimentaire dont il convient de rappeler qu'il qu'il était l'un des principes directeurs de la construction européenne dans les années 60 il vient en outre affaiblir notre balance commerciale agroalimentaire aujourd'hui encore excédentaire grâce aux céréales précisément et aux vins et spiritueux, sans oublier qu'il génère des transports par camions de céréales venant de zones de plus en plus éloignées, il y a un site des prairies pour y planter et planté encore ce qui, sur un plan écologique n'est pas très satisfaisant, enfin, il entraîne une augmentation du prix des céréales que les éleveurs du mal à supporter, ils n'osent pas, il que ce système intéresse un nombre grandissant d'investisseurs et offre à de nombreux agriculteurs et des possibilités de reconversion totale ou partielle, pour autant, il fonctionne selon un modèle économique artificielle car subventionné, alors même qu'il peut porter atteinte à environnement au regard de ce constat, pouvez-vous éclairer la représentation nationale sur la stratégie de l'État dans le domaine de la méthanisation. Merci beaucoup, madame la présidente, messieurs et mesdames les sénatrices et et sénateur Monsieur le le sénateur misons vous m'interrogez sur un sujet extrêmement important qui est celui de la méthanisation, c'est un sujet extrêmement important et votre question n'a bien montré parce que cette cette méthanisation à la fois une opportunité mais aussi une menace pour le monde agricole évidemment cette méthanisation, elle est source d'opportunité d'opportunités, vous l'avez dit économique d'opportunités environnementale également cette méthanisation fait partie notamment des objectifs de développement des énergies renouvelables et donc à ce titre au regard de ces opportunités, moi je défends la méthanisation, je pense que la méthanisation doit être soutenu dans notre pays, mais il faut le faire avec raison pourquoi il faut le faire avec raison parce que, en même temps cette méthanisation, elle peut être source de danger, de côté, pardon, tous les contrôles sur les infrastructures, au titre des polices environnementales mais peut-être un danger pour le monde agricole lui-même lorsque les productions agricoles viennent à être en compétition les unes par rapport aux autres, on dit souvent qu'en Allemagne l'élevage laitier a disparu du fait de la méthanisation, c'est probablement excessif, mais c'est un signal qu'il nous faut prendre en compte ce que je veux dire par là c'est que ma position, celle du gouvernement, a toujours été de dire oui, il faut défendre la méthanisation soutenir la méthanisation et c'est très bien de développer la méthanisation, je suis en soutien de cette méthanisation, mais en même temps, il faut créer le cadre propice à un développement de la méthanisation qui préserve ses équilibres agricole, pour ne pour ne parler que d'eux, alors c'est ce que nous avons fait avec la réglementation du 7 juillet 2016, c'est ce que propose d'ailleurs l'excellent rapport sénatorial fait par le président s'annonce sur le sujet une piste parmi d'autres, moi je pense que tout projet de méthanisation par exemple sur un territoire devrait faire l'objet, a minima, ni l'obstacle de la profession agricole par exemple des chambres d'agriculture, cela pourrait être une bonne piste à suivre. Merci. Monsieur Millon, vous avez 18 secondes. Merci monsieur le ministre, vous avez parlé d'une méthanisation raisonné que je partage, mais sur le terrain concrètement en mesure pas les dispositions que vous avez prises pour on en arriver là, on a le sentiment en tout cas dans le département de la Moselle que chacun fait comme il veut et que le 1er qui démarre à raison, donc, je crois, je pense qu'il vous devrez vous engager à prendre des à faire des mesures de contrôle pour but de vérifier ce qui se passe. Merci, cher collègue, la parole est à Madame Christine touché pour la question orale numéro 1943 Ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, je souhaiterais vous parler des forêts publiques et en particulier de la place que vous comptez confiée à l'Office national des forêts dans votre stratégie forestière nationale en effet les enjeux écologiques et environnementaux requiert d'adapter sans tarder la forêt au changement climatique d'initier leur renouvellement pour protéger la biodiversité, de répondre aux besoins de la société en produits de bois en s'appuyant surtout sur les écosystèmes naturels comme vous, a alerté à ce sujet une tribune de plus de 600 scientifiques et acteurs du secteur forestier dans le Journal du dimanche, à ce titre, le volet forestier du plan de relance a été doté de 200 millions d'euros pour les 2 prochaines années, destiné aux propriétaires forestiers, publics et privés, témoignant de l'engagement du gouvernement en faveur de la préservation de notre Patrimoine forestier et nous le saluons cependant l'ONF continuent de vivre une décrue de ses effectifs et une diminution constante de son budget, qui demeure largement déficitaire ainsi le projet de contrat entre l'État et l'ONF pour la période 2021 2025, nourri de vives inquiétudes pour son avenir, notamment en match en matière de stratégie sylvicoles et de réduction de la masse salariale et d'autant plus encore depuis l'annulation pourtant compréhensible attendu la contribution des communes forestières comment serait-elle sera-t-elle d'ailleurs compenser ce désengagement de l'État a pour conséquence la disparition des emplois de terrain comme nous le constatons dans l'Eure et de la perte d'un service d'accompagnement de proximité des communes. Alors indispensable effectivement pour l'exercice de leur mission d'intérêt général et de gestion de qualité de leur Patrimoine forestier, ces mesures ont véritablement des conséquences contradictoires avec les ambitions affichées du gouvernement et les exigences de la lutte contre le changement climatique, en conséquence, alors que les assises du bois ont été lancés seront clôturées fin janvier, nous souhaiterions être rassurés et en savoir un peu plus sur vos intentions quant à l'avenir de l'ONF et de ses missions pour la gestion durable de nos massifs communaux et domaniaux. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Julien Denormandie Ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. Merci beaucoup, madame la présidente, madame la sénatrice plus chez je dois vous dire que, en responsabilité, c'est à la fois. Assumer d'investir, mais ceci est à la fois assumer de régler les difficultés lorsqu'il y a des difficultés. L'ONF est un office incroyablement précieux dans notre pays, incroyablement précieux, je connais bien cette maison, je suis moi même ingénieur forestier et je peux vous dire et vous le savez, sur le terrain, à quel point l'ONF pour les forêts domaniales pour les forêts communales est un un office absolument précieux je salue toutes celles et ceux qui travaillent, dire que l'État se désengage des politiques forestières, alors même que l'État, vous l'avez dit dans votre question, investi plus de 200 millions dans le plan de relance, mais au final, ce sera 800 millions avec France 2030, me paraît un tout petit peu caricaturale, en tout cas pas conforme à la réalité, alors oui, l'État investit massivement dans cette politique sylvicole avec une politique, une vision qui est très clair : il forêt ça se protège, mais ça se cultive aussi et une forêt d'ailleurs aussi un atout sociétal pour beaucoup de nos concitoyens, qu'il faut développer et en même temps l'État en responsabilité doit faire face aux difficultés que traverse l'office et pour faire face à ces difficultés, nous faisons 2 choses : oui, nous avons conclu ce contrat État ONF oui, nous avons dit que nous ne ferons pas cette demande de contribution supplémentaire aux communes forestières, hé oui, nous avons dit à l'ONF dans le cas de ce contrat, d'une part, il faut que l'ONF contribue à elle-même, à faire face aux difficultés qu'elle a aujourd'hui c'est la trajectoire à la fois en termes RH et en terme managérial, mais également l'État doit investir beaucoup plus dans l'ONF, songez que dans la dernière loi de finances, qui n'a pas été discutée. Ici, c'est 60 millions d'euros supplémentaires mobilisés sur 3 ans pour soutenir l'ONF, ces 30 millions d'euros alloués en 21 à l'ONF pour. Situation des forêts domaniales et c'est plusieurs dizaines de millions d'euros que l'ONF dans l'ONF bénéficie d'enquête du plan France relance donc oui, nous continuerons à investir massivement dans cet office. Merci, Monsieur le Ministre, je rappelle qu'il faut rester dans ce temps sur avant vous, finalement, c'est un quart d'heure depuis le le début avec une question en moins, puisque le le sénateur n'était pas là, donc les collègues comme les doivent respecter leur temps pour que les autres puissent aussi y travailler, la parole est à madame Chantal de scène pour la question orale numéro 1987 au ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. Madame la présidente, monsieur le ministre, ma question porte sur les phénomènes d'augmentation des prix qui impacte fortement notre agriculture ces augmentations concernent le coût des carburants pour les véhicules, celui du gaz pour les opérations de séchage quant à la fin des pénuries autorise ses approvisionnements, mais aussi l'inflation des engrais azotés qui est supérieure à 300 % au cours des derniers mois, le sujet a été largement évoquée pour ce qui concerne le coût des énergies au travers de ma question, je souhaite attirer votre attention sur les marges de manoeuvre offertes concernant le coût des engrais à travers la levée des droits à l'importation et des taxes douanières anti-dumping selon la Chambre d'agriculture de mon département, l'Eure-et-Loir, l'impact économique actuel des augmentations de prix est évalué à 40000 euros par exploitation, monsieur le Ministre, au regard des difficultés que rencontrent nos agriculteurs, quelles sont les intentions du gouvernement afin de ne pas les laisser face à de nouvelles difficultés qui ne manquerait pas d'avoir des répercussions sur le pouvoir d'achat des consommateurs et sur notre compétitivité agricole, je vous remercie. Merci, la parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre de l'agriculture, de l'alimentation. Merci madame la présidente, madame la sénatrice de Seine plusieurs choses : d'abord cette crise des engrais, elle a un impact considérable sur la sécurité alimentaire mondiale et elle permet de rappeler à chacun que le rôle 1er de l'agriculture, c'est un rôle nourricier et que il y a une corrélation directe entre les engrais et la production alimentaire et donc c'est très important chez notamment saisi la FAO sur ce sujet il y a peu, parce que pour moi, c'est un sujet incroyablement stratégique 2ème élément, il y a 3 sujets il y a la question des coûts et comme vous l'avez dit dans votre question, la France a poussé continuer à pousser au niveau européen, la suspension de ce qu'on appelle des droits Ad Valorem j'ai initiée avant d'être président du Conseil, en tant que ministre de l'Agriculture, cette demande auprès de la Commission européenne, qui sont toujours ces sujets en cours de discussion avec elle 2ème point il y a un sujet de disponibilité nous avons organisé avec la filière avec les producteurs des voies et moyens pour s'assurer de la disponibilité en engrais, nous avons des unités de production, pas sur tout type d'ancrer je ne rentre pas dans le détail, mais nous avons des unités de production en France, à la différence d'ailleurs d'autres pays européens, et le 3ème sujet c'est un sujet de logistique parce qu'une fois qu'on a assuré la disponibilité, il faut s'assurer de la logistique avec des moments de tension et qu'il a aussi fait l'objet d'un suivi très particulier de mon ministère de celui des transports, en lien avec les professionnels, donc oui, il faut se battre sur ces 3 fronts : la question du prix avec cette taxation dites Ad Valorem au niveau européen, cette question de la disponibilité et cette question du transport logistique ce sujet il est fondamental parce que dans le contexte actuel, les Anglais ne l'oublions jamais, il faut évidemment d'avoir une utilisation raisonnée mais il ne faut jamais perdre de vue que ces engrais ces engrais sont le mot, le moment où la prendre, se nourrit et que vous avez une corrélation directe entre les engrais et le niveau de production. Madame de scène, vous avez 51 secondes. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, je sais que vous connaissez parfaitement toutes ces questions effectivement l'engrais est important, il nourrit la plante et ça garantit sa qualité mais alors que l'agriculture connaît, quel que soit le type d'agriculture d'ailleurs des difficultés et des passes difficiles, comment je réitère ma question : comment on peut intervenir pour que les coûts seront soit plus abordables parce qu'en fait on est sur des marchés parallèles, le marché des céréales et le marché des engrais et de la et de l'azote en particulier qui fait que les écarts sont énormes et que les les agriculteurs appréhende l'année à venir et la récolte à venir parce que, autant ils ont plus pour certains bénéficier de de de prix conséquence cette année, on n'est pas on n'est pas assuré que l'année prochaine on ne connaissent les mêmes conditions, je vous remercie. Merci, la parole est à Monsieur Daniel Chassain pour la question orale, numéro 2001 au Ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs années la filière bois, souffre de l'arrivée massive d'acheteurs étrangers, notamment chinois et, en plus des spéculateurs, ainsi le prix d'achat du bois atteint des sommets et les volumes disponible pour les séries françaises se raréfient, en conséquence, plusieurs secteurs industriels en aval, commence à donner des signes de tension, faute d'approvisionnement, j'ai pu échanger avec 2 séries de mon département qui font le même constat et partagent un même manque de visibilité limitant pour l'avenir, leur capacité d'investissement, selon les chiffres aux douaniers chinois, les exportations du chef français vers la Chine ont augmenté de 42 % celle des résines de 66 % seul en 2021 alors que de nombreux pays producteurs de bois, membre de l'Union européenne, ou non, ont pris des mesures limitant son exportation sous une forme brute, la France se laisse un peu pillé malgré le Label UE contournée par les acheteurs chinois, devrons-nous attendre que la concurrence chinoise chinoise asphyxie nos petites séries et menace davantage notre filière française, monsieur le Ministre, en plus d'interdire l'export de bois brut la filière propose des solutions qui ne dépend que d'une volonté politique nationale la stricte application des règles phytosanitaires qui renchérirait le coût de l'export et l'obligation pour les exploitants forestiers individuel de choisir entre l'exonération de l'impôt sur le revenu issu de ses ventes et des aides Monsieur le Ministre : quelle stratégie suit le gouvernement pour assurer l'approvisionnement des séries françaises et maintenir la valeur ajoutée des emplois en France. la parole est à monsieur Julien Denormandie Ministre de l'agriculture, de l'alimentation. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur, chassant le sujet Les d'une importance cruciale, je peux vous dire qu'on est à pied d'oeuvre depuis de longs mois sur cette situation qui est une situation d'ailleurs assez ancienne, qu'on a connu dans d'autres essences comme l'essence il y a, il y a quelques années et qui aujourd'hui est absolument tragique dans la filière du chêne, c'est en plus une aberration, une aberration écologique, une aberration en termes de souveraineté, les exportations ont augmenté de 30 % sur les 10 premiers mois de l'année 2021, en revanche, dans votre question il y a une une une erreur factuelle, très peu de pays européens ont mis en place des dispositifs d'interdiction à l'export et d'ailleurs elle n'a pas marché dans ce contexte qu'est ce qu'on qu'est-ce qu'on doit faire en fait, on doit lutter contre des traders et des traders chinois qui malheureusement ne sont lit pas limitée par le cou et donc les propositions que vous faites à la fin ne voient ne vont pas forcément venir trouver une solution puisque la question est que ces personnes qu'on a en face ne sont pas limités par le coup à chaque fois, renchérissent encore plus fortement, il y a 3 choses qu'on suit la première s'est porté au niveau européen, parce que c'est au niveau européen ces sujets d'de l'interdiction d'exportation, c'est ce que ce qu'on a fait depuis maintenant de, de, de longs mois et on continue à pousser ce sujet-là, le 2ème élément, c'est qu'à très court terme, on sait quelle est la solution à très court terme ces de massifier le recours au la pour les forêts publiques domaniales et communales toute vente de chaîne et soit sous le Label UE soit sous forme de contractualisation et donc on règle le problème comme cela immense difficulté c'est ce qu'on fait dans la forêt publique il faut maintenant le faire dans la forêt privée mais la question c'est : comment vous arrivez à convaincre les propriétaires forestiers de passer à ce Label, UE, sachant que vous avez cette liberté constitutionnelle ou un propriétaire est libre de l'utilisation de son bien, enfin le 3ème volet c'est d'avoir recours dans le futur encore plus massivement à la contractualisation qui est très important, mais à très court terme, c'est le sujet du Label UE qu'on pousse avec force. Monsieur le ministre Monsieur Chassaing, vous avez 10 secondes. Madame la présidente, donc comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, le poids de la forêt française devrait permettre à la France de peser au niveau européen afin de de mettre de mettre en place ces règles limitant l'export du bois brut. Si Monsieur Chassaing, la parole est à Monsieur Jean-Jacques Michaux pour la question orale, numéro 2000 34 au ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. Madame la présidente, monsieur le ministre, ma question concerne un problème récurrent dans mon département, auquel il est désormais urgent d'apporter des réponses claires, je veux parler de l'incertitude juridique qui entoure le statut des chiens de protection de troupeaux, en effet, dans nos territoires et particulièrement en Ariège, cette question du statut des chiens de protection soulève de nombreuses interrogations depuis plusieurs mois, ces chiens sont au coeur de nombreux conflits d'usage, qu'il s'agisse de poursuites à l'encontre d'éleveurs dans les chiens ont attaqué les promeneur ou randonneur ou des plaintes de voisinage pour cause de bruit occasionné par ces chiens, quand ils ne sont plus dans les estives la multiplication de ces conflits maudit de plus en plus les formes de gendarmerie et entraîne de nombreuses interrogations et inquiétudes chez les éleveurs, les bergers et les élus, pourtant, il s'agit bien là d'un comportement tout à fait légitime d'un chien de protection au travail dans l'Euro le 1er et d'éloigner tout intrus approchant le troupeau, comme vous le savez, les chiens de protection constitue une des mesures, aidé par l'État dans le cadre de la coexistence avec des grands prédateurs que sont l'ours ou le loup, ils sont l'un des éléments constitutifs de l'indemnisation des éleveurs en cas d'attaques du prédateur, les éleveurs antennes qui, s'il était amené à changer leurs pratiques pour s'adapter à ces nouveaux risques et mis en place la protection exigés par l'État, il est donc évident que cette contrainte ne peut se traduire in fine et pour eux par des difficultés supplémentaires : il semble donc nécessaire qu'une sécurité juridique spécifique aux chiens de protection soit apportées à ces éleveurs dans leur activité d'élevage et de pastoralisme aussi Monsieur le ministre, le gouvernement entend-il donner un statut juridique particulier aux chiens de protection afin de protéger juridiquement les procès le verre et les bergers, je vous remercie. Merci, la parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. Merci beaucoup, madame la présidente, monsieur le sénateur Jean-Jacques Michaux je partage totalement votre question sur la question du statut juridique des chiens de troupeaux, nous avons d'ores et déjà engagé la réflexion depuis la mi-2011 sur la question de la révision de ce statut, à la fois dans le cadre de la détention et de l'utilisation de ces chiens de 2 de 2 troupeaux afin que les travaux puissent se terminer le plus rapidement possible courant 2022, c'est d'ailleurs quelque chose que le président de la République a annoncé dès la fin de de l'été 2021 lorsqu'il en discuter avec les jeunes s'agriculteurs et les travaux sont précisément en ce moment donc je partage totalement ce que ce que vous avez dit j'en profite d'ailleurs pour dire que ces travaux, il part, il porte sur la gestion des chiens de troupeaux dont on connaît toutes les conséquences que cela peut avoir pour l'éleveur au quotidien mais il porte aussi sur un 2ème, sujet qui je crois très important, c'est la question du du comptage des loups parce que. Oui, il faut réussir à faire une cohabitation mais la cohabitation, elle ne peut pas se faire sur le dos de l'éleveur et qu'à chaque fois qu'il y a une attaque, c'est un drame pour l'éleveur, il faut avoir une approche très humaine de ces sujets, moi j'ai jamais été de ceux qui disent : vous inquiétez pas, au pire des cas, il y aura une indemnisation non, le travail de l'éleveur, c'est tout autre chose, c'est son Patrimoine des animaux qu'ils aient qu'il élève et donc il faut avoir cette approche humaine et dans cette approche humaine il y a évidemment la question des prélèvements, mais ces prélèvements si vous n'êtes pas d'accord sur le constat, c'est-à-, dire combien y a-t-il de loup sur le territoire, c'est quand même sacrément difficile ensuite de vous mettre d'accord sur la solution, c'est à dire de combien de loups, doit-on prélever combien de loups, doit-on prélever et donc cette revue du comptage avec là aussi une grande méthodologie, elle est également en course, ces 2 chantiers, chiens de troupeaux et comptages qui ont été ouverts par le président de la République le 1er ministre il y a quelques mois et qui sont en cours en ce moment. Merci, Monsieur le Ministre, la parole est à monsieur Bernard buis en remplacement de Monsieur Georges Patient, auteur de la question et donc la question numéro 2 1054 qui est posée au ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser mon collègue Georges Patient qui m'a demandé de vous poser sa question, il a en effet dû rejoigne la Guyane pour accueillir le ministre des Outre-Mer en visite depuis hier sur son territoire, monsieur le Ministre des acteurs de la filière bois, premier employeur privé de Guyane après le secteur spatial sont inquiets, très inquiets pour leur propre survie c'est un secteur classé par le gouvernement parmi les axes prioritaires de développement du territoire comme le confirme, et le président de la République lors de son déplacement en Guyane, en octobre 2017, cela s'est traduit par l'adoption en 2018 d'un programme régional de la forêt et du bois PR FB dans lesquels il est prévu de multiplier par 3 les volumes de bois d'oeuvre issues de la forêt naturelle le volume annuel de grumes extrait passerait ainsi à 210000 à l'horizon 2030, or la particularité de la forêt guyanaise et la certification éco-responsable son exploitation pratique unique dans la région amazonienne imposant aux exploitants forestiers de s'enfoncer toujours plus profondément en forêt pour trouver les arbres exploitable, ils utilisent pour cela les pistes dans l'ONF a la responsabilité, en tant que gestionnaire du domaine forestier permanent, le Pr FB prévoit un investissement de 5 millions d'euros par an jusqu'en 2000 29 pour la création de nouvelles pistes afin d'offrir à l'exploitation de nouveaux massifs forestiers en l'ONF viennent d'annoncer, limiter l'investissement annuel pour les pistes à 2 millions d'euros à partir de cette année quant 3 millions d'euros, jusqu'à présent, l'Union européenne rembourse pourtant à 100 % ses travaux via le Feder, pourquoi ne pas en profiter, certes il faut les préfinancer le temps du déblocage des fonds européens environ 3 ans, cela représente une avance de 15 millions d'euros, ces investissements conditionne la survie de la filière au lieu d'un triplement des volumes extraits sans les nouvelles pistes les volumes vont au contraire chuter en raison de l'épuisement de la ressource dans les massifs aujourd'hui accessible manière de matières premières, toute la filière sera touché au risque de la voir disparaître, c'est pourquoi, Monsieur le Ministre, le gouvernement doit autoriser et l'ONF Guyane après financer les 3 années d'avance de trésorerie. Merci, la parole est à monsieur Julien Denormandie Ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. Merci beaucoup, madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le, le sénateur Buy, permettez-moi de de saluer votre collègue Georges Patient, dont je connais l'engagement sur cette question des forêts guyanaises à l'évidence, comme vous l'avez dit dans la votre question, nous devons d'être extrêmement vigilants sur ce niveau d'investissements dans la création d'une desserte forestière précisément pour les raisons que votre collègue Georges Patient dans dans sa question, alors c'est vrai que les pouvoirs publics finance depuis plusieurs années, jusqu'à 100 % de ses investissements pour la création d'une desserte, notamment dans le cadre de l'apport des fonds européens, c'est-à-dire le Feader vous l'avez dit aussi, même si ces investissements sont financés à 100 % l'ONF doit en faire l'avance de trésorerie jusqu'au remboursement et, tout en devant assurer l'entretien des dessertes en place, les acteurs économiques de guyen sollicitent que le le montant d'investissement qui n'a pas pu être réalisée en 2021 puisse être en 2022 afin de rattraper le retard et donnant ainsi plus de visibilité, de lisibilité conformément à votre demande ou, plus précisément celle du de votre collègue Georges Patient que vous transmettez aujourd'hui et je tiens à vous dire en en retour que le gouvernement a bien entendu cette demande et que les crédits du programme 149 du ministère ont été réévalués en 2022 pour assurer la contrepartie la contrepartie pardon national nécessaires au financement du fait d'erreur et permettre ainsi à l'ONF de réaliser ces investissements en cohérence avec le programme régional de la forêt et du bois, le montant prévisionnel des investissements de création de pistes prévue en 2022 devrait donc pouvoir atteindre plus de 4 millions d'euros, répondant ainsi à votre question, et l'ONF ajustera donc l'enveloppe allouée à la direction territoriale de Guyane. Pour les crédits nécessaires afin de faire ce préfinancement et de faire le financement, comme je viens de vous l'indiquer, Monsieur le Sénateur. Merci, la parole est à monsieur Alain Cazabonne pour la question orale numéro 1620 au Ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. Merci madame la présidente, mes chers collègues, monsieur le Ministre, l'Office français de la biodiversité, considèrent les produits de la mer non commercialisés comme des déchets, on compte parmi les 10 produits les moules de soutien ou encore des coquilles vides d'huîtres vides, ces produits, rejetés à la mer viennent de la mer sans avoir subi aucune altération modifications ainsi, il s'agit de produits naturels remis dans leur milieu naturel en outre les procédures ont été établies dans les délibérations de comités régionaux conchylicole afin de limiter les rejets Anta, source de nuisances visuelles et durant la période estivale olfactive, surtout à cause d'utilisation d'agricole, la demande est celle-ci : est ce qu'il peut y avoir une clarification sur ces produits de la mer non commercialisés, afin que ces derniers ne soient plus considérés comme des déchets. la parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur Alain Cazabonne alors en fait la réponse à votre question est relative à la nature de de ce dont on parle, et notamment des différents mollusques bivalves pour les appeler comme il se doit, dont on on. On doit prendre en considération les caractéristiques, c'est-à-dire que les moules, par exemple, destinés à la consommation humaine qui sont récoltés dans les élevages, font l'objet de de de règles spécifiques au type d'un d'un règlement, le fameux règlement 853 que les professionnels connaissent, et donc à ce titre, elles ont un statut de denrées alimentaires et de produits d'origine animale, elles sont. Pour certaines, notamment les moules sous taille, exclu de la consommation humaine par les producteurs pour des raisons essentiellement commerciales et il découle de ce procès, ce que ces moules sous taille, ce sont des sous-produits animaux de catégorie 3. Du fait des caractéristiques qui qui sont ceux que celle que je viens de dire, et donc lorsque vous êtes face un sous-produit animal de catégorie 3 le règlement en question établi les règles sanitaires applicables. à la gestion de ces sous-produits, là je parle des moules sous taille c'est-à-dire de de mollusques bivalves qui reste vivant, ce n'est pas la coquille vide et là ils sont considérés comme des sous-produits animaux de catégorie 3 pour un ensemble d'raisons évidemment des des raisons sanitaires, que tout le monde connaît bien et donc. Les producteurs, dans ce cas-là, pour les moules sous taille ont l'obligation de trier dit s'identifier et de prendre en charge, comme le dit ce règlement, en revanche, l'application directe dans les sols de ces sous-produits n'est pas explicitement prévu par le règlement comme un usage possible mais ce qui n'est pas le cas en en revanche des coquilles d'huîtres, quant à elle, qui et plus largement des coquilles de mollusques qui vide son corps mou ou chèque. Non pas le statut de sous-produits animaux et dans ce cas-là, peuvent être utilisés comme vous venez de le dire, monsieur le sénateur. Si Monsieur Casabonne vous avez une minute et 10 secondes. Monsieur le Ministre, merci, j'ai 50 60 % de de réponses positives, ce que je comprends tout à fait parce que c'est vrai que les coquilles non non aucun présente aucun danger et je pense que pour les agriculteurs pour les agriculteurs pour les conchyliculteurs, c'est quand même déjà importante de pouvoir séparer cette partie, ça leur fera moins de tracas administratifs et même de surcoût merci. Merci, la parole est à monsieur Bernard buis ce cette fois-ci c'est pour vous la question orale, numéro 2 1056 transmise au ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, l'obligation de débroussaillement d'une et d'arbustes d'arbres ou végétaux divers débordant d'une propriété privée sur la voie publique incombe au propriétaire, nous le savons tous mais ce sujet reste problématique est régulièrement soulevé auprès des maires par leurs administrés en effet le code forestier impose à ses propriétaires, d'assurer l'entretien non seulement de leur propriété mais aussi des parcelles non bâties qui jouxte leur propriété sous certaines conditions, ainsi, l'article L 131 tiré 11 permet au préfet de rendre obligatoire le débroussaillement sur les fonds voisin jusqu'à une distance de 50 mètres de l'habitation, le propriétaire négligent d'intérêt non bâti peut de cette façon faire porter la responsabilité sur ses voisins, propriétaire d'une construction en parallèle le code général des collectivités locales, dans son article L. 22 permet aux maires de mettre en demeure le propriétaire négligent d'exécuter les travaux d'entretien de sa parcelle à proximité d'habitations dans la distance de 50 mètres, bref l'articulation de ces 2 textes rend difficilement compréhensible, les obligations qui pèsent à chacune des parties, c'est pourquoi monsieur le ministre, je vous interroge afin d'apporter une nécessaire clarification tant pour les mères que pour les propriétaires concernés. Merci, la parole est à monsieur Julien Denormandie Ministre de l'Agriculture et de l'alimentation. Merci beaucoup, madame la présidente, monsieur le sénateur, je vois bien là dans votre question, la précision qui vous caractérise, j'avoue que moi-même quand j'ai vu votre question, je n'étais pas forcément conscients de ce distinguo qui, somme toute, mérite d'être précisé pour qu'il soit compris par tous, peut-être même un jour mieux explicitées par le pouvoir législateurs législateur que vous êtes en fait, il faut distinguer parce que votre question pour faire samedi, parfois ça incombe au maire se débroussaillement et parfois ça incombe au préfet dès lors que ça n'ait pas fait par le propriétaire. Lui-même, en fait, il faut distinguer les territoires, c'est-à-dire que dans les territoires réputé particulièrement exposés aux risques d'incendie de forêt hostile des articles L 132 et elles sont 33 tiré hein et votre département, par exemple, la Drôme en fait partie alors c'est aux maires d'assurer le contrôle de l'exécution des obligations de égal de débroussaillement, en revanche, en dehors de ces territoires, le code près Forissier prévoit dans l'article que vous avez mentionné le L 131 tiré 11 la possibilité pour le préfet de ponctuellement prescrire des obligations légales de débroussaillement équivalente après appréciation du risque incendie. Et d'ailleurs, cette disposition aux mains des préfets et peut-être pas suffisamment connus et mériterait d'être mieux explicitées vis-à-vis de l'ensemble des interlocuteurs de de terrain, voilà ce que je pouvais vous dire Monsieur le le sénateur dans le distinguo pour essayer de répondre à mon tour, de la manière la plus précise possible à votre question. Merci, monsieur, vous avez 45 secondes. Non, juste pour remercier Monsieur le Ministre, de ces précisions, qui je pense, était très importante parce que de nombreux maires nous interroge régulièrement, donc ça ferait passer votre réponse merci beaucoup. Merci beaucoup, la parole est à Monsieur, Cédric Perrin pour la question orale numéro 1905, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Merci madame la présidente, madame la ministre, je me doute que vous n'est pas suivi de près, mais multiple, questions et alertent sur cette problématique c'est bien normal, le dossier que j'aborde aujourd'hui est un dossier technique qui relève du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, je me quand je me contenterai donc de rappeler les faits connus par la ministre gourou en 2 mots : depuis depuis plus de 2 ans maintenant, je ne cesse d'interpeller le gouvernement sur les conséquences financières de l'implantation de l'hôpital Nord Franche Comté sur la petite commune de trêve non ces frais de gestion de l'état civil, dont bien évidemment exploser plusieurs options ont été envisagées, mais aucune à ce jour n'a été retenue ou même expérimenté en dépit de promesses du cabinet de Madame Gourault devant le maire de la commune, le 7 mai 2021 pour trouver une solution, quelques mois plus tard le 15 octobre cette fois en l'absence du maire, les conseillers de la ministre plaidait en faveur d'un accord que je savais déjà impossibles entre les parties prenantes, cet insecte occasions que nous avons bien compris qu'il fallait que l'on se débrouille, si je ne peux obtenir l'aide du gouvernement sur le fond de ce dossier, je souhaite a minima recueillir son interprétation juridique sur l'article suivant 223 21 23 21 pardon tiré 5 du code général des collectivités territoriales, dispose qu'à défaut d'accord entre les communes concernées sur leur contribution respective ou de création d'un service commun chargé de l'exercice de ses compétences, la contribution de chaque commune a fixé par le représentant de l'État dans le département du siège de l'établissement public de santé, ma question est donc simple : à Madame la Ministre, dans quelles conditions s'organise le déclenchement de cette procédure de fixation de la contribution de chaque commune par le représentant de l'État, dès lors que les communes concernées, constate qu'un accord entre elle et définitivement impossibles, je vous remercie. Merci, la parole est Madame, Nadia et pour ministre délégué chargé de la ville pour 2 minutes. Madame la présidente, monsieur le sénateur, Cédric Perrin je crois que la ministre, Jacqueline Gourault a déjà eu l'occasion de le rappeler dans sa réponse du 14 avril dernier à votre question, qui portait sur la charge financière des missions d'état civil par la commune de trêve, non du fait de la présence de l'hôpital Nord Franche Comté, la loi prévoit un mécanisme de compensation au profit de la commune d'implantation de l'établissement public de santé, comportant une maternité, ce mécanisme est une contribution financière des communes extérieures qui repose sur la différence entre la les naissances comptabiliser le nombre d'habitants de la commune sur le territoire où se situe l'établissement, elle s'applique à toutes les communes ayant plus d'1 % de naissance ou de décès dans cet établissement, nous pourrions faire bouger ces seuils nous n'y sommes pas défavorables sur le principe, mais il faudra ouvrir ce chantier avec l'AMF car il y a des conséquences pour des centaines de communes en outre la création d'un service commun entre l'EPCI et ses communes afin de mutualiser les missions d'état civil et d'en répartir les coûts avaient été évoquée et je regrette que cette solution à la main des acteurs locaux n'ait pu aboutir faute d'accord entre les communes, cependant, la commune dispose d'autres leviers pour financer, c'est en 1er lieu elle peut solliciter son EPCI afin qu'il augmente le montant de contribution de compensation sa surface financière pourrait lui permettent de procéder à Sète hausse sans nuire à son équilibre budgétaire et pour participer au financement d'un équipement structurant de son territoire, en second lieu, la commune peut solliciter le conseil départemental pour qu'il tienne compte de sa spécificité dans les critères qu'le détermine pour répartir le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ou le Fonds départemental de de péréquation des DMTO par exemple, le département de de Belfort versent chaque année 1,8 millions d'euros du FDP été TP aux communes, la loi prévoit que l'importance des charges et des communes doit être un critère et le gouvernement n'envisage pas, comme vous le demander de rétablir les taxes funéraire sur les convois, les illuminations et les crémations supprimée par la loi de finances pour 2021, en revanche, si le vocable des taxes vous même en réalité les redevances aucune. L'immersion de la fait obstacle merci madame la Ministre, comme vous venez d'arriver, je vais vous faire tout de suite à nos petit rappel à l'ordre à ne pas dépasser, parce que si vous prenez 10 secondes à chaque question, vous voyez, ça, ça prend beaucoup de temps, monsieur Perrin, vous avez 14 secondes. Une fois de plus, je n'obtient pas gain de cause et vous continuez à expliquer aux collectivités qu'elles doivent prendre en charge ce que l'État ne souhaite plus faire aujourd'hui la taxe funéraire a été supprimé, tout a été supprimé et aujourd'hui d'une collectivité de 2000 habitants doit prendre en charge la totalité de la naissance d'une d'un d'un département de près de 150000 habitants, ce qui est évidemment. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur François Calvet pour la question orale numéro 1983 la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Merci madame la présidente, madame la ministre je souhaite attirer votre attention sur les conséquences du transfert obligatoire de la compétence voirie aux communautés urbaines prévue par la loi, notre pour la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée métropole le 1er janvier 2016, la communauté d'agglomération de Perpignan Méditerranée est devenue la communauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole regroupant 30 ceci communes précédemment et en conformité avec la loi notre la compétence voirie étaient exercées par les communes, s'agissant d'une compétences optionnelles ou facultatives des communautés d'agglomération mais depuis le 1er janvier 2016 demandes de gestion cohabitent : d'une part au moyen de convention de gestion qui permettent aux communes de continuer à gérer directement la compétence voirie, le personnel est restée communal, les Budgets de fonctionnement et d'investissement sont communaux et gérée par la commune et les marchés travaux sont initiés, suivi par la commune, la communauté urbaine rembourse tous les ans les frais de fonctionnement et d'investissement aux Communes ce mode de gestion constituer une tolérance juridique transitoire destinée à permettre aux communautés urbaines, de mettre en oeuvre le transfert de la compétence voirie, d'autre part, au moyen de 2 pôles territoriaux regroupant chacun des communes qui lui ont transféré le personnel ainsi que la gestion financière et opérationnelle de la compétence voirie cette dernière organisation territorialisée des concentrés permet à la communauté urbaine de gérer directement la compétence voirie tout en préservant les besoins de proximité, il niera inhérents à cette compétence ce double système de fonctionnement à la satisfaction de tous, je souhaite savoir si une telle régime peut perdurer ou devenir moment de de gestion de la compétence voirie par les communautés urbaines et dans le cas inverse, ce qu'il convient de faire merci. Merci, la parole est à Madame, Nadia et ministre délégué chargé de la ville. Monsieur le sénateur François Calvet depuis la loi Chevènement de 99 l'avoir est une compétence obligatoire des communautés urbaines et au 1er janvier 2016, la communauté d'agglomération Perpignan-Méditerranée a demandé à devenir communauté urbaine, ce qui implique implique une intégration intercommunale supérieur, il est donc elle est donc compétente en matière de voirie, depuis lors, les recours aux conventions de gestion que vous mentionnez également nommé convention de prestation de services sont prévues par les dispositions de l'article que vous avez cité du CG toutefois ces conventions ne doivent pas constituer un moyen pour un EPCI à fiscalité propre de rétrocéder aux communes des compétences qui lui ont été transférés par le législateur, nous partageons avec vous l'impératif de répondre au besoin de proximité dans l'exercice de cette compétence en associant, en particulier les maires des outils sont à la disposition des acteurs locaux tout d'abord, le pacte de gouvernance peut prévoir les conditions dans lesquelles l'EPCI à fiscalité propre peut déléguer aux maires d'une commune, membre de l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant d'infrastructures de bâtiments communautaires le maire dispose donc d'une autorité fonctionnelle sur les services concernés les réunions de la conférence des maires favorise également le dialogue entre entre ces collectivités et lorsqu'un EPCI à fiscalité propre forme une commission, il faut aussi prévoir la participation des conseillers municipaux des communes membres selon des modalités qui le détermine ensuite, il est possible, comme vous l'évoquez de prévoir une organisation déconcentrée des services intercommunaux, chargé de la voirie, la plupart des grandes intercommunalités l'ont mis en place afin de répondre en proximité aux besoins des populations dans des délais adaptés aux travaux d'entretien courants enfin dans le cadre de son pouvoir de police générale que lui confère notamment la responsabilité d'assurer la sûreté et la commodité du passage sur les voies publiques, le maire peut intervenir pour assurer la sécurité de la population, c'est une détérioration de la voirie exigeait une intervention urgente. Merci. La parole est à monsieur Alain Milon la question orale, numéro 2021, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Oui merci madame la présidente, madame la ministre, depuis le 1er janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, la fameuse Gemapi, est une compétence confiée aux intercours par les lois de décentralisation de 2014 et 2015 progressivement cette compétence est passé d'une réglementation sur l'ouvrage digue à une réglementation sur le système d'endiguement actuellement plus d'une centaine de ses structures en France est confrontée à cette impossibilité de trouver un assureur Groupama qui intervenait jusqu'à présent ne soumissionnent plus ce désengagement est particulièrement préjudiciable pour ces établissements, qui exerce une compétence majeure pour la protection de nos concitoyens, notamment par endettement, en vertu du principe qui veut que l'État soit son propre assureur, la prise en charge de ces risques ne posait pas des difficultés avant le transfert de cette compétence depuis le transfert, la question se pose avec une réelle réelle acuité consultez le bureau central de tarification n'a pu apporter de solutions à cette problématique dans la mesure où sa structure de droit public peuvent être leur propre assureur, or la plupart de ces structures intercommunales, n'ont pas la capacité financière pour assurer ses risques en auto-assurance, eu égard à l'ampleur du risque à couvrir, alors même que l'année inondations un des probabilités d'occurrence de plus en plus importante leur capacité financière s'avère insuffisante pour assumer la couverture de ces risques en cas de survenance d'une catastrophe naturelle, outre les difficultés majeures engendrés par cette situation, il est pour le moins paradoxal de constater cette frilosité des compagnies d'assurance à remplir leur mission envers des structures qui oeuvrent à la prévention des risques, avec pour objectif de limiter les dégâts occasionnés, ce qui induit Rey une diminution des remboursements. Quelles mesures donc Madame Elis, entendez-vous prendre pour résoudre cette situation et permettre à ces structures d'exercer leurs compétences dans des conditions satisfaisantes, tant du point de vue financier que d'amis en cours sécurité des populations concernées. Merci, la parole est à Madame, Nadia et ministre délégué chargé de la ville. Monsieur le sénateur Alain Milon, comme vous le savez la compétence Gemapi dont les missions sont confiées sont définis pardon par le code de l'environnement, on est a été confiée par le législateur à titre obligatoire aux EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018, les syndicats de rivière qui exerçaient tout ou partie des missions Gemapi avant cette date, ont pu se maintenir, via le mécanisme de la représentation substitution toutefois, ces structures sont invités à fusionner ou à étendre leur périmètre pour atteindre une taille hydro-graphique est cohérente avec la gestion efficace du grand cycle de l'eau leur transformation en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau, les pages notamment, il non en établissements publics territoriaux de bassin et tu en ce sens, vivement encouragé ce changement d'échelle leur permettrait de constituer les provisions nécessaires pour régler les coûts engendrés par d'éventuels sinistres dans le cadre du système de l'auto-assurance, la nouvelle organisation de la Gemapi n'alourdit pas la responsabilité du gestionnaire d'ouvrage qui ne peut être engagée dès lors qu'on a qu'ont été respecté les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception leur exploitation et à leur entretien par ailleurs et surtout la Gemapi peut-être financé par les ressources non affectées du budget général et ou par une taxe facultative plafonné un équivalent de 40 euros par habitant et par an, et dédié exclusivement à la prise en charge de cette compétence en cas de transfert de tout ou partie de la compétence Gemapi un syndicat mixte l'EPCI à fiscalité Ports propres peut lever la taxe Gemapi pour financer sa contribution statutaire, le projet de loi 3DS en cours de discussion au Parlement prévoit par ailleurs la possibilité pour les EPTB à titre expérimental de lever des contributions afin de financer la Gemapi enrichissant encore le dispositif actuel, enfin plusieurs dispositifs permettent de soutenir les collectivités dans leur rôle de prévention des risques naturels, c'est le cas notamment du fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds Barnier, même s'il varie, elle varie logiquement selon l'échelle de mutualisation choisit la capacité financière d'exercer la Gemapi est donc assurée. Oui, je vous n'avez pas répondu à la question est de la même histoire : je vous demande quels sont les assureurs qui pourrait assurer les syndicats et les collectivités territoriales, femme, je ne vous ai pas demandé de me refaire la loi que nous connaissons par coeur. Merci. La parole est à monsieur Jean-Yves Roux pour la question orale, numéro 2 1042 au secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, 2000 22 et tu n'étais pas une étape importante pour le concitoyen, c'est celle de la démilitarisation de nos services publics, c'est aussi celui du très haut débit pour tous avant un fibrage de l'ensemble du territoire prévue en 2025, dans les Alpes-de-Haute-Provence, malgré des besoins immenses les objectifs ne sont pas tenus, seuls 40 communes sur les 178 faisant partie de la Mel sont raccordés à la fibre et pas en totalité dans ces conditions, le télétravail pourtant préconisée en ce moment n'est pas possible la réservation en ligne du service de santé de vaccination non plus la continuité pédagogique et discontinue quant aux services publics en ligne dans nos communes, ils sont intermittents plus inquiétant, la qualité des records demain est à revoir un dépit d'une convention en bonne et due forme avalisée par arrêté en mai 2019 avec SFR Altice il s'avère que la réalité des travaux de raccordement est pour le moins folklorique des câbles trop tendu qui cède un des virages de route en montagne il y en a des lignes enfouies qui deviennent aérienne et inversement, des poteaux appartenant à l'opérateur historique eux aussi historique des boîtiers laisser ouvert de l'Open Beta, sans parler des conditions de sécurité au travail qui font peur, nos mères nous rapporte cerise sur le gâteau, être tenu à l'écart d'autorisation de voirie les plus élémentaires et constate des chantiers, un chantier et des et gages sauvage leurs questions et demandes de réparation, on appelle bien souvent que du silence hors du silence au mépris parfois à la marge est faible, je suis sûre, Madame la Ministre, que vous partagez notre colère parce que nous le constatons les moyens ont été mis sur la table comme jamais, y compris avec le plan de relance pourtant aujourd'hui dans notre département le fibrage avant ce peu et mal fait coûte de l'argent et beaucoup d'énergie à l'ensemble des collectivités, il y a matière à redresser la barre en ce moment puisqu'un autre à la ruralité de notre département ont besoin d'une preuve d'amour, Madame la Ministre que comptez-vous faire pour apaiser les tensions entre les différents protagonistes de la fibre ici SFR et Orange qui se renvoient la balle, comment allez-vous impulser une exigence de qualité. Si chaque fois merci je pense que Madame la Ministre, vous a quoi M. le ministre, vous avez la parole. Monsieur le sénateur Jean-Yves Roux, vous en êtes je crois enfin, convaincu que le gouvernement aujourd'hui accorde une priorité sur la couverture numérique dans nos territoires et le président de la République a fixé l'objectif de généralisation de l'accès à la fibre optique sur le territoire, à horizon 2025, en complément des initiatives privées et publiques, le gouvernement a offert la possibilité aux collectivités de faire appel aux opérateurs privés dans le cadre d'une procédure d'appel à manifestations d'engagements locaux pour déployer la fibre optique sur leurs fonds propres, le syndicat mixte ouvert sud THD associant votre département, celui des Hautes-Alpes et des Bouches-du-Rhône, ainsi que le conseil régional PACA a fait ce choix en 2018, les engagements de SFR acceptée par arrêté ministériel du 20 mai 2019 vise la couverture en fibre optique, des locaux de l'ensemble de la zone d'initiative publique initiale, soit près de 300000 locaux à horizon 2022, ces engagements sont opposables aux sous et soumis à sanctions de l'Arcep sur le fondement de l'article L. 33 tiré 13 du code des postes de D et des communications électroniques à l'échelle locale une convention cadre signé par les exécutifs de chaque collectivité territoriale et l'opérateur XP fibres et à laquelle l'État n'est pas partie prenante permet d'organiser les modalités de suivi des déploiements s'il se réjouit de la dynamique de déploiement de la fibre, le gouvernement est vigilant quant au respect par les opérateurs du cadre réglementaire et de la qualité des déploiements à ce titre, l'Arcep a annoncé fin novembre 2021, l'ouverture d'une enquête administrative sur expect fibres et ses filiales et à l'échelle des Alpes de Haute-Provence là une société est en lien permanent avec les collectivités territoriales et la préfecture, la présidente du conseil départemental et la préfète porte par ailleurs une attention spécifique aux bonnes conditions de déploiement de la fibre optique par HP xp fibres et elle co-présideront le 24 février prochain comité de concertation départementale. Merci, la parole est à monsieur Claude Kern pour la question orale numéro 1967 transmise au ministre de l'Intérieur. Merci madame la présidente, madame la ministre, je souhaiterais à terre, attirer votre attention sur les forêts funéraire, une forêt cinéraires, est un site d'inhumation d'urne biodégradable qui permet, dans le respect de la dignité due au corps humain de vivre le deuil différemment, en offrant une alternative plus économique et de prendre en compte d'autres facteurs, ce type d'inhumation intéresse de plus en plus de familles et de collectivités, ces nouveaux lieux de mémoire d'apaisement et de sérénité en pleine nature, trouvent tout leur sens dans le constat que beaucoup de cimetières sont actuellement saturés et nécessite des travaux d'agrandissement qui dans certains cas sont difficiles à réaliser par manque d'espace vice-disponible ce mode de sépulture existe déjà dans plusieurs pays en Europe, dont, parmi les plus proches, la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne, à titre d'exemple chez nos proches voisins du Bade Würtemberg, il existe des Budgets mais elle Hanoï ainsi à Reynaud cette pratique fonctionne parfaitement dans ce pays, interpellé par plusieurs collectivités de mon département notamment ne Villers Les Saverne et la somme Ayrault serait-il envisageable de modifier la législation française et d'autoriser cette alternative à la sépulture en cimetière pour répondre à une demande de plus en plus croissante. Merci, la parole est à Madame, Nadia et ministre délégué chargé de la ville.

relève de la compétence exclusive des communes et des EPCI ceci, on l'a vu là l'initiative de leur création, son propriétaire du site et en assure la gestion des emplacements sur le site itinéraire isolés

aménagé à cet effet, quant à la légalité, de créer un site cinéraires isolé dans une forêt, je ne peux vous donner une réponse de portée générale, un espace arboré ou forestiers peut théoriquement être envisagés pour l'implantation d'un site cinéraires isolé pour ces projets, comme pour les cimetières, il est nécessaire de se conformer au régime juridique applicable en l'état du droit qui permet de veiller au respect de la dignité des défunts et à la pérennité des sites choisis, le maire de la commune d'implantation doit également pouvoir y exercer pleinement ses pouvoirs de police spéciale en matière de funéraire de funérailles, pardon, enfin tout projet dit de forêt funéraire doit être appréhendé au regard du régime forestier régis par le code forestier dès lors que ce régime a été rendue applicable à la forêt aussi, aussi, il n'y a pas lieu de créer de statut de règles particulières à l'implantation de lieux de sépulture en forêt, plutôt qu'ailleurs. Merci. Si Monsieur K, mais vous avez 47 secondes. Merci madame la ministre, j'ai bien entendu vos explications que ça s'appelle site funéraires isolé ou forêt funéraire, malheureusement, il y a des communes qui ont tenté l'expérience, je veux citer la commune d'Arbas en Haute-Garonne et qui se heurtent après à des blocages administratifs du à des contradictions même des services de l'État, donc il faudrait peut-être accorder les violons dans ce dans ce service, et afin de faire bénéficier aux vos familles d'un mode de sépulture respectueux de l'environnement et des dernières volontés des défunts. merci, la parole est à Madame Agnès Canayer pour la question orale, numéro 2000 45 à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Merci madame la présidente, madame la ministre, donc les opérations de recensement oblige chaque année les communes a réalisé pour le compte de l'État, le comptage de leur population pour les grandes communes chaque année une partie de leur territoire et soumis à ces opérations de recensement pour les plus petites, elles doivent le réalisée tous les 5 ans, ces opérations des conséquences fortes pour les communes notamment puisqu'elles induisent le montant des subventions qui leur seront dévolus, vous n'êtes pas sans savoir que ces opérations de recensement qui commence dans 2 jours, ce fonds cette année dans un contexte épidémiologique particulier et, au plus fort du Pic du variant Omicron cela, bon j'ai générer des difficultés pour les communes, difficulté d'accéder chez les familles dans les maisons, notamment s'il y a des clusters, difficultés pour recruter les agents en ces périodes de contamination au nombre des agents communaux sont déjà eux-mêmes en arrêt de travail penser que cette opération de recensement pourront avoir lieu par voie numérique ou par voie des réseaux sociaux, hé bien mal connaître, madame la ministre, la vie communale, pourquoi ne pas avoir reporté ces opérations de recensement, pensez-vous pouvoir donner un délai supplémentaire aux communes pour faire face aux contraintes qui résulte de l'épidémie et enfin, comptez-vous indemnisées à juste hauteur ce coût lié à cette suggestion supplémentaire de la Covid pour les communes. Merci, la parole est à Madame, Nadia et ministre délégué chargé de la ville. l'importance toute l'importance que que constitue le recensement pour permettre notamment de dimensionner les services publics, que ce soit les crèches ou encore les transports et de déterminer la contribution de l'État au Budget de chaque commune, il est donc important qu'ils soient réalisés chaque année, l'Insee avait en raison du contexte sanitaire exceptionnel de 2020 et des restrictions en vigueur annoncé le report à 2022, et de l'enquête de recensement qui était prévue à l'origine, en janvier, février 2021 sauf à Mayotte où là ça a été effectivement réalisés cette année, la situation est différente, l'enquête de recensement, a pu être correctement préparé préparé à la fin de l'année 2021 et les restrictions liées à la crise sanitaire sont moindres que l'an dernier, notamment les déplacements ne sont pas limités par ailleurs l'accès à la vaccination permet de réduire fortement les risques sanitaires, les méthodes mises en oeuvre par l'Insee en 2021 pour calculer des populations légales en l'absence d'une enquête de recensement ne peuvent pas être reconduite, elle ne permettent pas de prendre en compte les mobilités résidentielles liée à la crise sanitaire et l'enquête de recensement de la population est une opération avec très peu de contact entre les agents recenseurs et les et et la population recensée, il est possible de répondre à l'enquête par Internet et pour les personnes qui souhaitent tout de même remplir un questionnaire papier, celui-ci ne se fait pas en présence de l'agent recenseur ce dernier passe uniquement pour déposer le formulaire ou reprendre le questionnaire les agents recenseurs n'ont donc pas besoin d'entrer dans les logements, compte tenu de ces dispositions, il n'y a pas, nous le pensons en tout cas de très gros risques sanitaires avec les éléments que je viens de vous communiquer le calendrier, a donc été maintenue et en cas de difficultés lors de la collecte, elles pourront toutefois demander un report de la date de fin de collecte que l'Insee examinera avec bienveillance. Oui merci madame la ministre, effectivement, on voit bien quand même que la crise épidémique continue dans des formes différentes, mais elles continuent, donc elle va rendent plus difficile quand même, la réalisation de cette opération de recensement et notamment les suggestions sur les communes, ça va changer des des coûts supplémentaires, parce qu'il va falloir trouver de nouveaux agents et ça va encore en générer générer des difficultés déjà que le remboursement de l'État des frais occasionnés par le recensement n'est pas à la hauteur du coût réel, je pense qu'il faudrait que l'État, cette fois-ci, prennent aussi en compte dans le cas de son quoi qu'il en coûte la véritable coût du recensement aujourd'hui pour les collectivités locales. Merci. Alors je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 14 heures 30 pour l'examen de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, la séance est suspendue.